J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération et, d'autre part, sur la proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire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 L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez aujourd'hui débattre de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale qui transpose en droit interne la directive européenne sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales des entreprises. Il s'agit d'un texte important, car il propose l'introduction dans notre législation d'un dispositif adapté et équilibré de protection du secret des affaires, attendu depuis de longues années. La proposition de loi qui vous est soumise est en effet le fruit d'une réflexion ancienne, très approfondie, au cours de laquelle toutes les parties prenantes auront été en mesure de s'exprimer. À l'échelon européen, tout d'abord, la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués a été adoptée en 2016, après la réalisation par la Commission européenne d'une large consultation publique et d'une solide étude d'impact. Les débats devant le Parlement européen ont permis de faire évoluer la proposition de directive afin que soient adoptées des mesures fortes de protection des droits fondamentaux. ensuite, de nombreux rapports et plusieurs initiatives parlementaires ont porté sur ce sujet au cours des quinze dernières années. Au-delà des clivages politiques, ces différentes initiatives ont mis en

Dans un premier avis, daté du 31 mars 2011, il avait souligné les obstacles juridiques auxquels se heurterait la mise en oeuvre d'une nouvelle infraction réprimant pénalement l'atteinte au secret des affaires. Saisi de l'examen de l'actuelle proposition de loi, qui comporte un dispositif civil de protection du secret des affaires, le Conseil d'État a rendu, le 15 mars dernier, un avis très éclairant sur l'opportunité pour le législateur national de se saisir des marges de manoeuvre offertes offertes par la directive afin, en particulier, de renforcer la protection accordée au secret sur le plan procédural devant les juridictions judiciaires ou administratives. Ainsi, contrairement à certaines opinions exprimées lors des débats devant l'Assemblée nationale, ce sont non pas l'opacité et le secret qui ont présidé à l'adoption de la directive puis au dépôt de la proposition de loi au Parlement, mais, bien au contraire, l'analyse économique, la réflexion juridique, la transparence et le débat d'idées. Vous ne l'ignorez pas, cette réforme est, depuis plusieurs années, très attendue des entreprises ; la protection des informations relevant du secret des affaires est évidemment essentielle pour nos acteurs économiques, pour encourager l'innovation et préserver les stratégies industrielles et commerciales. C'est par l'innovation ainsi protégée que seront créés les emplois attendus par nos concitoyens. L'enjeu est donc fort : il s'agit de lutter contre l'espionnage industriel et de garantir la compétitivité de nos entreprises au sein du marché intérieur. L'enjeu est aussi de renforcer l'attractivité de notre système juridique pour les investisseurs étrangers. Il faut permettre à l'ensemble des acteurs économiques d'empêcher, de faire cesser ou de réparer toute atteinte à un secret des affaires, en agissant, le cas échéant, très rapidement, devant un juge en requête ou en référé. Jusqu'à présent, notre législation ne comportait aucune définition de cette notion de secret des affaires, alors que celle-ci figure déjà dans de nombreux textes avec d'autres notions équivalentes telles que le secret industriel et commercial. La protection du secret des affaires reposait en France sur le droit commun de la responsabilité civile, qui est principalement d'origine jurisprudentielle. Enfin, à l'exception des actions en dommages et intérêts liées à des pratiques anticoncurrentielles, aucune règle écrite n'encadrait la protection du secret des affaires au cours des procédures judiciaires. La proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise permet indéniablement de répondre au besoin de sécurité juridique des acteurs économiques. Elle définit le secret des affaires et procède à une harmonisation, dans dans différents codes, de terminologies employées pour désigner les mêmes catégories d'information ; il s'agit là d'une réelle mesure de simplification.

Je souligne d'ailleurs ici la convergence de vues entre les commissions des lois des deux assemblées pour élargir la portée des mesures de protection du secret des affaires prévues à l'article 9 de la directive à l'ensemble des instances civiles, commerciales ou administratives. Comme l'a indiqué le Conseil d'État dans son avis du 15 mars dernier, cette solution présente « l'avantage d'harmoniser les procédures applicables devant le juge, quel que soit leur objet, ce qui va dans le sens d'une simplification et d'une plus grande lisibilité du droit ainsi que d'une protection plus effective du secret des affaires conforme aux objectifs de la directive Le texte adopté par l'Assemblée nationale me paraît reposer sur un équilibre satisfaisant entre, d'une part, la protection du secret des affaires et, d'autre part, le respect des principes fondamentaux de la procédure civile, au premier rang desquels se trouve le principe du contradictoire. Enfin- c'est d'une très grande importance -, la proposition de loi permet de poser des limites au droit à la protection du secret des affaires, puisque ce droit ne saurait être absolu. Il est en effet indispensable, dans une société démocratique, que certains secrets puissent être divulgués, dans un but d'intérêt général. Ces secrets peuvent être révélés par des journalistes exerçant leur liberté d'information. Ils peuvent être révélés pour l'exercice des droits des salariés au sein de l'entreprise. Ils peuvent également être divulgués par un lanceur d'alerte qui, au sens de la directive, révèle une faute, un acte illégal ou un comportement répréhensible. Les juridictions gardiennes des libertés individuelles feront la balance des intérêts en présence en veillant notamment à ce qu'aucune condamnation ne puisse intervenir à l'encontre d'un lanceur d'alerte au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II. Nous aurons l'occasion, au cours des débats, d'aborder plus particulièrement la protection des lanceurs d'alerte, puisque votre commission des lois

Si l'introduction dans notre droit d'une définition du secret des affaires et d'un encadrement normatif de sa protection suscite de nombreuses inquiétudes ou critiques- vous avez pu les lire dans différents journaux je crois que les débats devant la représentation nationale sont essentiels pour expliquer aux Français les réels enjeux de la proposition de loi, faire ainsi oeuvre de pédagogie et, par voie de conséquence, apaiser les craintes. l'affirme de nouveau devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, la protection du secret des affaires en Europe et en France, qui n'est pas nouvelle, sera désormais mieux encadrée, au bénéfice de tous, et cette protection ne conduira à aucune restriction des droits fondamentaux. Je veux à ce titre remercier M. le sénateur Christophe-André Frassa, votre rapporteur au nom de la commission des lois. La qualité de nos échanges a été réelle sur ce texte important, et vos travaux, monsieur le rapporteur, auront indéniablement contribué à enrichir de façon très constructive le débat, dans la continuité de l'important travail réalisé par M. le député Raphaël Gauvain. Même si, Même si, sur certains sujets, nos points de vue divergent, je sais que nous partageons le même objectif de lisibilité et d'intelligibilité de la norme, de transposition fidèle de la directive et de recherche d'un équilibre satisfaisant entre différents intérêts en présence, comme en témoignent les amendements que vous avez proposés et qui ont été adoptés par la commission des lois. Permettez-moi d'évoquer plus particulièrement deux évolutions importantes apportées au texte adopté par l'Assemblée nationale. Tout d'abord, votre commission des lois a souhaité supprimer la disposition relative à l'amende civile pour recours abusif introduite par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Rappelons que cette mesure mesure visait à prévenir et, le cas échéant, à sanctionner les procédures abusives qui, en la matière, peuvent porter une atteinte particulièrement forte à l'exercice de ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression.

Les sanctions prévues par le droit commun sont-elles suffisamment dissuasives au regard de l'atteinte qui peut être portée, notamment, à l'encontre des journalistes et des lanceurs d'alerte exposés à des demandes volontairement excessives en dommages et intérêts ? Vous nous demandez également si les sanctions prévues sont ou non disproportionnées au regard du principe constitutionnel de proportionnalité des peines, qui s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition. On peut estimer que la mesure adoptée par l'Assemblée nationale permet, au contraire, d'apporter une réponse équilibrée aux risques dénoncés de procédures abusives ayant pour seul objectif d'empêcher la révélation de faits intéressant l'intérêt général.

Votre surprise n'a d'égale que ma propre assurance ... Ensuite, votre commission des lois a souhaité introduire au sein du code pénal un nouveau délit de « détournement d'une information économique protégée afin de sanctionner d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros toute atteinte à un secret des affaires commise dans le but d'en retirer un avantage exclusivement économique. Je comprends, bien entendu, votre légitime préoccupation d'introduire dans notre droit un dispositif suffisamment complet et efficace de protection du secret des affaires, dans un contexte de concurrence exacerbée entre les acteurs économiques. Toutefois, je crois qu'il n'est pas nécessaire, à cette fin, de compléter l'arsenal juridique qui résultera de la transposition de la directive. Au-delà des réelles difficultés juridiques soulignées par le Conseil d'État dans son avis du 31 mars 2011, et qui demeurent pertinentes, l'opportunité de surtransposer la directive en créant une nouvelle sanction pénale ne me paraît pas démontrée. D'une part, le dispositif civil résultant de cette transposition répondra au besoin des entreprises de pouvoir agir rapidement en justice afin de prévenir toute atteinte imminente ou de faire cesser toute atteinte illicite au secret des affaires, mais permettra aussi d'obtenir la réparation intégrale part, il est d'ores et déjà possible de sanctionner pénalement une entreprise qui s'approprie frauduleusement le secret des affaires d'une entreprise concurrente, soit dans le but d'en tirer profit, soit dans un but de déstabilisation. Des faits d'atteinte à un secret des affaires peuvent notamment être qualifiés de vol, d'abus de confiance ou d'extraction de données dans un système informatisé de données. Je pense par conséquent que, dès lors que l'insuffisance du droit pénal n'a pas été démontrée, Pour l'ensemble de ces raisons, je présenterai au nom du Gouvernement un amendement revenant sur l'article instaurant ce nouveau délit réprimant l'atteinte à un secret des affaires. Je présenterai également quelques amendements destinés à apporter au texte qui vous est soumis des corrections techniques qui me paraissent utiles. Je ne doute pas un instant de la qualité des discussions qui vont suivre. Je souhaite de nouveau remercier tout particulièrement M. le sénateur Christophe-André Frassa et les membres de la commission des lois pour le travail accompli. Je remercie aussi l'ensemble des membres de votre assemblée qui contribueront à nos débats afin d'introduire, dans notre droit, un dispositif complet, efficace et équilibré de protection des informations relevant du secret des affaires. Mes chers Mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer, en votre nom, la présence dans notre tribune d'honneur d'une délégation de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc, conduite par M. Abdessamad Kayouh, président du groupe d'amitié Maroc-France de la Chambre des Conseillers. La délégation est accompagnée par M. Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et président du groupe d'amitié sénatorial France-Maroc, et par des membres de son groupe. Le Maroc est engagé, depuis de nombreuses années, dans une politique ambitieuse de réformes- politiques, économiques, sociales -, notamment dans le domaine de l'environnement. Le Maroc a d'ailleurs accueilli avec succès en 2016 la COP 22 à Marrakech, à la suite des accords de Paris. Cette visite s'inscrit dans ce cadre,

français des entreprises, pouvant résulter de la confrontation entre le système juridique français et certains systèmes juridiques étrangers, en particulier anglo-saxons. De ces travaux, il ressortait notamment

Ces constats demeurent malheureusement valables. Toutefois, la présente proposition de loi devrait permettre de surmonter la première de ces difficultés majeures pour les entreprises françaises, connue depuis longtemps, dans des conditions d'égalité avec les autres entreprises de l'Union européenne. Je déplore qu'il ait fallu attendre la transposition d'une directive- qui plus est, à la fin du délai de transposition, la directive datant de juin 2016 -pour se doter enfin d'un régime de protection légale du secret des affaires en droit français. ailleurs relever ce paradoxe : alors qu'il a fallu attendre des années pour que notre pays puisse se doter d'un tel régime, nous devons aujourd'hui examiner dans des délais extrêmement contraints le texte qui concrétise cette longue attente.

dans l'information de la société civile. Un équilibre a été trouvé entre les exigences également légitimes de protection du secret des affaires des entreprises et d'information tant des salariés que des citoyens. La directive considère que « les secrets d'affaires sont l'une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus couramment utilisées par les entreprises, et, en même temps, ils sont les moins protégés par le cadre juridique existant de l'Union contre l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite par d'autres parties Dans certains domaines bien circonscrits, le droit français ne connaît que la notion traditionnelle de secret industriel et commercial et, dans de rares cas, la notion de secret des affaires. Quelques dispositifs épars et sectoriels ne constituent pas une protection générale et transversale contre l'obtention illicite de secrets d'entreprises non légalement protégés. Le constat est clair : il manque à la législation française un dispositif général et transversal de protection du secret des affaires garantissant une vraie protection des informations confidentielles détenues par les entreprises françaises. Le constat de la carence du droit français en matière de protection du secret des affaires est connu depuis longtemps, de sorte que les initiatives n'ont pas manqué ; aucune, toutefois, n'a pu aboutir jusqu'à présent. En novembre 2011, notre ancien collègue député Bernard Carayon, que j'ai entendu en audition, déposa une proposition de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires, qui fut adoptée en janvier 2012 par l'Assemblée nationale, juste avant la fin de la législature. Cette proposition de loi ne comportait qu'une dimension pénale visant à dissuader plus fortement la captation illicite de secrets d'entreprises par leurs concurrentes. Controversé dans les milieux économiques, ce texte est demeuré sans suite devant notre assemblée. En juillet 2014, quelques mois après la présentation de la proposition de directive, notre ancien collègue député Jean-Jacques Urvoas, alors président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, déposa une proposition de loi relative à la protection du secret des affaires, comportant à la fois un volet civil et un volet pénal. Quelques mois plus tard, les dispositions de cette proposition de loi furent introduites par l'Assemblée nationale, en première lecture, au stade de la commission, dans la dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, avant d'en être retirées dès la séance, au vu de la vive controverse médiatique qu'elles suscitèrent. Je relève que le contexte n'est plus le même aujourd'hui, avec l'obligation de transposition d'une directive européenne. Venons-en maintenant au texte qui nous est soumis. Sur mon initiative, votre commission des lois a adopté 24 amendements visant à assurer la conformité de la proposition de loi à la directive, à préciser et à clarifier les procédures judiciaires mises en place par le texte, dérogation au secret des affaires, aux journalistes, aux lanceurs d'alerte et aux représentants des salariés, et à créer un délit de détournement à des fins économiques d'une information protégée au titre du secret des affaires, afin de mieux sanctionner les atteintes frauduleuses aux intérêts des entreprises françaises par des concurrents. Tirant les conséquences des modifications et ajouts apportés au texte initial de la proposition de loi par l'Assemblée nationale puis par elle-même, votre commission l'a renommée « proposition de loi relative à la protection du secret des affaires ». Votre commission a veillé à la conformité de la proposition de loi à la directive. En particulier, elle a distingué, à l'instar de la directive, les notions de « détenteur légitime » et d'« obtention licite » du secret des affaires, alors que la proposition de loi confond ces deux notions, en retenant le critère du contrôle sur le secret pour définir le détenteur légitime. Elle a aussi précisé que l'ingénierie inverse constituait un mode licite d'obtention, mais sous réserve de stipulations contractuelles interdisant ou limitant l'obtention du secret. Elle a également retenu une formulation plus conforme à la directive de l'obtention illicite d'un secret, caractérisée notamment par un accès non autorisé à un support contenant le secret, et non par une interdiction

loi énonce que le secret « n'est pas protégé », rédaction soulevant de nombreuses interrogations quant à sa portée juridique effective. Par conséquent, votre commission a préféré indiquer que le secret n'est pas opposable en cas d'instance relative à une atteinte au secret des affaires, en précisant clairement qu'il reste protégé ultérieurement dans les cas où il n'a pas été divulgué au public par un journaliste

Elle a ainsi expressément prévu les règles de prescription en matière d'action civile pour atteinte au secret des affaires. Elle a harmonisé, par cohérence, les règles d'évaluation des préjudices avec celles qui sont prévues en matière de propriété industrielle et de contrefaçon. Elle a également précisé et clarifié les dispositions relatives à la protection du En outre, votre commission a veillé à la constitutionnalité du texte en supprimant le mécanisme d'amende civile prévu en cas de procédure abusive engagée pour atteinte au secret des affaires, en raison de sa contrariété avec le principe de proportionnalité des peines. D'ailleurs, compte de la pratique judiciaire, les juges n'auraient jamais appliqué cette sanction civile. Votre commission a approuvé les exceptions au secret des affaires ouvertes au bénéfice des journalistes, des lanceurs d'alerte et des représentants des salariés, au nom de la liberté d'expression et d'information, tout en clarifiant la portée juridique des dispositions proposées par le texte. L'équilibre doit être conservé entre les exigences également légitimes de protection du secret des affaires des entreprises et de libre information des citoyens. En ce qui concerne les journalistes, votre commission a, à l'issue d'un débat, adopté le texte sans modification, considérant que l'amendement que j'avais présenté pour clarifier le texte pouvait susciter des incompréhensions. En ce qui concerne les lanceurs d'alerte, votre commission a distingué plus clairement l'existence d'un double régime d'alerte, celui qui est issu de la directive et celui qui a été instauré en 2016 par le législateur français. La transposition de la directive ne doit en effet pas conduire à la remise en cause du régime français, plus protecteur des lanceurs d'alerte. Les incriminations pénales existantes ne permettent pas de prendre correctement en compte toutes les hypothèses de violation du secret des affaires à des fins purement économiques. En conséquence, votre commission a créé un délit de détournement d'une information économique protégée consistant à obtenir, à utiliser ou à divulguer de façon illicite une information protégée par le secret des affaires en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d'en retirer un avantage de nature exclusivement économique. Les peines encourues seraient les mêmes que pour l'abus de confiance, c'est-à-dire trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. La conformité du dispositif au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines serait assurée par la définition précise de ses éléments matériel- le fait de contourner sciemment les mesures de protection mises en place par le détenteur légitime du secret -et intentionnel- le but d'en retirer un avantage de nature exclusivement économique. Les journalistes, les lanceurs d'alerte et les représentants des salariés seraient clairement exclus du champ de ce délit, puisqu'il vise l'obtention d'un avantage de nature exclusivement économique. Il s'agit ainsi de renforcer la portée dissuasive de la nouvelle législation française en matière de secret des affaires, à l'égard notamment de certains intérêts étrangers qui pourraient considérer que la simple action civile ne représente pas une réelle menace de sanction en cas d'obtention illicite d'une information confidentielle d'entreprise protégée par la loi.

Madame la ministre,

cette directive par le Parlement européen et le Sénat, avec une résolution que vous avez adoptée le 11 juillet 2014, approuvant les orientations retenues par la Commission.

veux évoquer le nécessaire équilibre entre secret des affaires et liberté d'information Notre rapport a ciblé quelques dispositions à ajuster, mais, sur le fond,

Je pense en particulier, sur ce point, à l'insertion d'un renvoi à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, bien sûr, à la définition des éléments d'ordre

Si notre assemblée a une totale latitude législative dans la limite d'une transposition et n'est donc en rien tenue de s'aligner sur les positions du Parlement européen ou de l'Assemblée nationale, comme le souligne fréquemment le président de notre commission des lois,

quel exploit ! Nous nous devions, en cet instant, de le souligner. « Exploit », c'est ainsi qu'il convient de qualifier la présentation, devant notre Haute Assemblée, de cette proposition de loi venue du Palais-Bourbon.

deux mois montre en main, avec une commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale se réunissant avant même que Conseil d'État ne rende son avis. C'est un exploit au vu des différentes tentatives pour inscrire le secret des affaires dans notre droit positif. un exploit au vu de la difficulté que rencontre la doctrine à définir précisément le secret des affaires. C'est un exploit, enfin, si l'on compare ce texte avec la proposition de loi portant sur la revalorisation des retraites agricoles, déposée par notre groupe, qui, malgré le soutien d'une très large majorité du Sénat, est encore en instance, alors que, dans le même temps, on nous invite à discuter d'un texte déposé le 19 février dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale. Hélas ! Sur la forme, cette proposition de loi est un bien utile pour éviter d'en passer par un projet de loi, lequel aurait nécessité une étude d'impact et aurait possiblement bien plus médiatisé le contenu de la directive européenne relative au secret des affaires. ! Cette absence, sur un texte aux conséquences aussi lourdes et incertaines sur la liberté de la presse et la liberté d'information, est en soi suffisante, à nos yeux, pour refuser de le voter. À cela s'ajoute le caractère risible de l'argument du vide juridique, qui expliquerait l'impérieuse nécessité de transposer ces dispositions dans le droit français, lequel serait, nous dit-on, totalement dépourvu de garanties de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle des secrets de fabrication. Dès lors que son double caractère inutile et hasardeux est acté, se pose la question de ce qu'est cette directive, qui a suscité plusieurs pétitions rassemblant, rappelons-le, plus de 550 000 signataires,

Il a été largement démontré que cette directive a été écrite sous la dictée des multinationales elles-mêmes. Nous ne reviendrons pas sur les problèmes posés par la comitologie bruxelloise et par le fléau que constitue le au niveau européen, fût-il encadré et déclaré. Nous pensons véritablement que ce texte, du point de vue du droit, est aux limites du conflit d'intérêts, éclairant d'un jour nouveau la conception de la « société civile » dans ce « nouveau monde ». À cet égard, il n'est pas inutile de revenir sur le processus législatif européen qui commence en 2013, dans la tourmente des « Panama Papers » ou encore des Luxleaks. Que fait alors la Commission européenne ? Elle ne propose ni plus ni moins que d'accorder la priorité à la protection du secret des affaires, notion au demeurant assez floue- elle l'est toujours aujourd'hui. À moins que le caractère « secret » de certaines affaires n'agisse précisément comme une sorte de tautologie, en vertu de laquelle les affaires sont secrètes parce qu'elles le sont ... Encore une fois, la Commission européenne a fait la preuve de sa grande capacité d'écoute et de compréhension de certains milieux d'affaires, dans une Europe dont les peuples s'interrogent de plus en plus sur la direction prise par la construction européenne elle-même. Sur le fond, cette proposition de loi sur le secret des affaires tend clairement à aller à contre-courant du sens de l'histoire.

La transparence s'impose partout comme une évidence, comme une nécessité démocratique essentielle dans nos sociétés. Mais ce mouvement s'arrêterait aux portes de l'entreprise. Cela est regrettable, pour ne pas dire inacceptable. De plus, l'un des points nodaux de la proposition de loi qui nous est soumise est d'arguer que le droit français serait dépourvu de protection du secret des affaires. Toutefois, en l'absence d'étude d'impact, il est impossible d'en avoir la certitude. Au reste, le renvoi à l'expertise européenne n'est pas acceptable, tout comme l'impossibilité d'en prévoir les effets juridiques. Les parlements nationaux ne peuvent sous-traiter cette étape essentielle du processus législatif. L'absence d'étude d'impact, tout anodine qu'elle puisse paraître, agit comme le révélateur de ce passage en force que l'on souhaite nous imposer avec l'adoption de ce texte. Relisons ce que disait l'auteur et rapporteur de la proposition de loi, M. Raphaël Gauvain : « Pourquoi protéger le secret des affaires ? Cette proposition de loi intervient pour combler un vide juridique : en France, la protection du secret des affaires relève pour l'essentiel de l'application jurisprudentielle des règles de droit commun de la responsabilité civile. Pourtant, de nombreux pays, parmi lesquels nos concurrents économiques, et en tout premier lieu les États-Unis, disposent depuis longtemps d'un arsenal législatif performant en la matière pour défendre leurs entreprises. » Un vide juridique ? Je crois pourtant savoir que nous sommes pourvus d'un droit de la propriété intellectuelle depuis un certain temps, et que celui-ci couvre, entre autres, la protection des marques, brevets, dessins, modèles et autres processus de fabrication, base du patrimoine immatériel de nos entreprises On peut même se demander, à la lecture de ces propos, si l'auteur de la proposition de loi sait que les services douaniers agissent depuis des décennies contre la contrefaçon en remontant les filières de production de produits parfois dangereux pour la santé.

que la volonté de faire primer le droit des affaires et, au sein de celui-ci, le secret des affaires sur toute autre considération. Protection de la liberté de l'information ? Texte équilibré ? Protection des lanceurs d'alerte et respect des libertés syndicales ? Comment dire ? ... Si nous ne savons toujours pas ce qu'est le secret des affaires- nous y reviendrons avec un cas d'espèce -, il est certain qu'un syndicaliste allemand pourra échanger en toute sécurité juridique avec ses collègues français ou belges du même groupe industriel à la condition expresse d'avoir prouvé qu'il ne mettait pas en péril le secret des affaires.

du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice. » Dans le cas contraire, engagera-t-on une procédure de licenciement pour faute lourde ? Prenons désormais un dernier exemple. La proposition de loi définit le secret des affaires comme toute information revêtant « une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de dit, une information commerciale donnée est couverte par le secret des affaires au motif qu'elle est secrète. La valeur de l'information, pour plus de précision, est d'ailleurs considérée comme effective ou potentielle, ce qui laisse imaginer on ne sait trop quoi ... Mes chers collègues, souhaitons bon courage aux juges

qu'il s'agirait de protéger des fichiers de clients ou de fournisseurs, des méthodes et des stratégies commerciales, des informations sur les coûts et les prix, les projets de développement, les sinistres ou encore les études de marché. Il y aurait donc urgence à couvrir du secret des affaires la réalité peu enviable de circuits d'approvisionnement conduisant vers les pays à bas coût salarial, à donner vertu aux méthodes de marketing les plus éculées, à laisser passer le jeu sur les prix de transfert et la possible vente à perte, à permettre la pratique des marges arrière ou encore du chantage permanent auprès des fournisseurs. Voilà sans doute une conception fort intéressante de l'économie par le prisme de ce secret des affaires, qui ne correspond nullement à l'intérêt général, mais qui satisfait plus sûrement quelques intérêts économiques et financiers bien particuliers, ainsi que leurs obligés avocats. Au nom de la transparence et du débat démocratique, je ne peux qu'inviter le Sénat à voter cette motion tendant à opposer la question préalable. Y a-t-il

moyen d'une proposition de loi, donc sans étude d'impact ; délai d'à peine deux semaines entre l'adoption en séance par l'Assemblée nationale et le passage en commission au Sénat ; examen quelques semaines seulement avant l'expiration du délai de transposition -, je souhaite mettre l'accent sur un point : l'adoption de la question préalable entraînerait le rejet du texte.

qui permettra une approche commune, globale. Il permet ensuite une articulation avec les autres droits fondamentaux, ce qui est nouveau.

chers collègues, pour la commission des affaires européennes, il est exact qu'il n'y a pas de surtransposition. Nous sommes dans l'épure de la directive. Toutefois, comme la directive le prévoit,

Il est vrai que les délais d'examen qui nous ont été imposés sont contraints. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera certainement pas la dernière

Le scrutin est ouvert.

la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, dite « secrets d'affaires », ayant pour but d'harmoniser la notion de secret des affaires, doit être transposée dans notre droit interne avant le 9 juin 2018. cette raison, une proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 19 février dernier, par les membres du groupe La République En Marche, et la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement. L'objectif est triple : mettre la France au niveau de protection des entreprises étrangères, offrir un cadre juridique européen commun et prévenir l'espionnage économique ou le « pillage » ou la divulgation des innovations à des concurrents. Il est ici question des brevets, des secrets de fabrication et, surtout, des données économiques de nos entreprises à l'heure du tout numérique. La directive a posé trois critères pour qualifier une information relevant du secret d'affaires ne pas être facilement accessible à des personnes extérieures à l'entreprise ; revêtir une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ; faire l'objet de mesures de protection raisonnables de la part de l'entreprise. Cette définition est reprise par le présent texte, qui prévoit également que les entreprises victimes de vols d'informations pourront ester en justice. Toute la difficulté de telles dispositions réside dans la manière de conjuguer la légitime protection du secret des affaires de nos entreprises et le respect des libertés fondamentales, telles que la liberté d'informer la société civile, dont les journalistes, les lanceurs d'alerte ou encore les représentants des salariés doivent pouvoir user. Les inquiétudes formulées par ces derniers ont, me semble-t-il, été entendues par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, qui a prévu un certain nombre de garde-fous non négligeables. En effet, le texte sorti de l'Assemblée nationale dispose que le secret des affaires ne peut s'appliquer lorsqu'il s'agit d'« exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse ». Ainsi, les entreprises ne pourraient se prévaloir du dispositif de la présente proposition de loi pour bloquer la publication d'une enquête ou réclamer des dommages et intérêts à un journal. il convient de rappeler que, en l'état actuel du droit, et avant même la transposition de la directive, des actions en justice sont d'ores et déjà engagées à l'encontre d'organes de presse. J'en veux pour preuve la très récente décision : cette enseigne a obtenu gain de cause pour faire retirer un article de l'hebdomadaire faisant état de ses difficultés financières- étant précisé qu'appel a été interjeté

Enfin, la proposition de loi organisait une troisième exception au secret des affaires pour les salariés obtenant des informations internes sur leur entreprise et les transmettant à leurs représentants, tels que les délégués syndicaux, si leur divulgation est « nécessaire » à l'exercice des fonctions dudit dudit représentant. En définitive, en intégrant le secret des affaires dans notre droit, fidèlement et dans les délais de la directive, il n'est pas question de porter atteinte à la liberté d'informer. Je comprends les craintes exprimées, mais le texte sorti de l'Assemblée nationale était parvenu à trouver un juste équilibre. Au lieu de chercher à hiérarchiser et, du même coup, à opposer les principes fondamentaux, il nous appartient, en tant que législateur, de réussir à les articuler les uns avec les autres.

Notre groupe a déposé un certain nombre d'amendements visant, notamment, à rétablir l'amende civile contre les procédures dilatoires ou abusives et à supprimer l'infraction pénale spéciale réprimant la violation du secret des affaires créée par la commission, que je juge superfétatoire. Nous conditionnerons notre vote à leur adoption ou, à tout le moins, à la présence de gages d'équilibre et de proportionnalité indispensables. La

nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre d'une proposition de loi visant à transposer la directive européenne du 8 juin 2016 relative au secret des affaires, dont le délai de transposition court jusqu'au 9 juin prochain. L'objectif de cette directive est, selon son exposé des motifs, de « mettre en place, au niveau de l'Union, des règles pour rapprocher les droits des États membres de façon à garantir qu'il y ait des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes dans le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires Il s'agit là d'un pas dans la bonne direction. Si les brevets et le savoir-faire technique brevetable sont depuis longtemps connus et reconnus comme des enjeux majeurs de la compétitivité de nos entreprises, les savoir-faire et informations commerciales n'en sont pas moins importants, en particulier au moment où les services constituent une part croissante de l'économie française. Les savoir-faire techniques et commerciaux représentent ensemble un capital intellectuel essentiel à une économie qui se veut une économie du savoir. Ne pas protéger ce capital, c'est laisser la porte ouverte à la concurrence déloyale et à l'effritement des atouts de nos entreprises. Or l'Europe a déjà pris du retard sur ses partenaires, notamment les États-Unis, qui ont adopté, dès 1979, une loi sur la protection des secrets commerciaux. C'est à ce titre que l'Union européenne s'est donné comme objectif, dans sa stratégie UE 2020, d'assurer une protection unifiée de la propriété intellectuelle, notamment de certains de ses aspects complémentaires, dont le secret des affaires. Cette protection passe par une harmonisation, à l'échelle de l'Europe, de la définition des secrets des affaires et la garantie qu'existe, dans chaque État membre, au moins une procédure au civil permettant de protéger ces informations sensibles. En France, le retard est tout particulièrement marqué : la notion même de « secret des affaires » ne dispose pas de définition unifiée dans notre droit. La loi dite « de blocage » du 26 juillet 1968 punissait, par exemple, les atteintes à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts économiques essentiels de la France. Or le droit de la régulation et de la concurrence, mais aussi les réalités économiques ont beaucoup évolué depuis lors. Il est donc devenu essentiel de moderniser l'outil juridique français et européen. Des initiatives prises par le passé dans ce sens, en particulier celle de notre collègue député Bernard Carayon en 2011, n'ont jusqu'ici pas abouti. Durant l'élaboration et la discussion de la directive et de la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui, une autre question a surgi, celle de la conciliation entre le secret des affaires et les activités d'information du public et de protection de l'intérêt général. Cette question ne concerne pas seulement les journalistes, mais aussi les lanceurs d'alerte. Il n'est pas possible d'ignorer leur contribution à l'intérêt général, comme l'ont illustré les « Panama papers ». Aussi le législateur européen s'est-il efforcé d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la protection des secrets des affaires et la sauvegarde des libertés journalistiques et de l'intérêt général. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, cette proposition de loi transpose la directive au sein d'un nouveau titre du livre premier du code de commerce consacré au secret des affaires.

Il s'agit de l'information qui, sans être généralement connue ou aisément accessible, revêt une valeur économique effective ou potentielle du fait même de son caractère secret et fait l'objet par son détenteur légitime de mesures de protection « raisonnables Puis, ce texte distingue les détenteurs légitimes, les personnes obtenant connaissance du secret des affaires de manière licite et les obtentions et divulgations illicites. dernières feraient l'objet d'un certain nombre d'exceptions destinées à garantir la capacité d'action des autorités de contrôle et de régulation, mais aussi à protéger l'activité des journalistes, des représentants des salariés et des lanceurs d'alerte. Le secret des affaires n'est alors pas opposable. À cet égard, le texte procède à une articulation bienvenue du secret des affaires avec la loi du 9 décembre 2016 relative à la protection des lanceurs d'alerte. La proposition de loi comprend également un certain nombre de dispositions permettant au juge civil de prévenir, faire cesser et réparer les atteintes au secret des affaires. Le juge et d'autres personnes pourront alors avoir accès au secret, mais demeureront tenus à la confidentialité. Enfin, le dernier article de la proposition de loi harmonise la terminologie utilisée par les textes français en matière de secret des affaires. Ce texte aura donc le mérite d'offrir de bonnes bases à la protection des secrets commerciaux et du savoir-faire commercial dans notre pays. La commission des lois et son rapporteur, mon éminent collègue Christophe-André Frassa, ont mené un travail d'amélioration que je tiens à saluer. Ils ont rendu la transposition plus fidèle à la directive et ont renforcé son impact sur notre compétitivité. Ainsi, le détenteur légitime d'un secret et ceux qui seront appelés à en prendre connaissance de manière licite seront désormais mieux distingués. Par ailleurs, le nouveau délit pénal d'espionnage économique, instauré à l'article 1, permettra de sanctionner spécifiquement les atteintes les plus déloyales à nos intérêts économiques et à ceux de nos entreprises. Malgré les apports indéniables à notre compétitivité que fournira cette proposition de loi, je tenais à regretter la méthode utilisée pour faire aboutir ce texte.

de loi. De l'aveu même des députés l'ayant portée, la proposition de loi initiale a été largement rédigée par la Chancellerie. Cette situation a privé le Parlement du bénéfice d'une étude d'impact approfondie, qui aurait pourtant été très utile dans ce domaine crucial pour la compétitivité de la France.

de notre rapporteur et des sénateurs qui ont été en première ligne sur ce texte, notamment mes collègues Jacques Bigot et Jean-Yves Leconte. Toutefois, au-delà même de la procédure accélérée, c'est le choix d'une proposition de loi qui pose question. On sait que des velléités de réforme, sur ce thème, avaient été éteintes lors des débats sur la loi Macron. On aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement aujourd'hui aux commandes du pays comprenne la charge lourde pesant sur ce texte.

Lundi dernier, une manifestation a rassemblé journalistes et lanceurs d'alerte, place de la République. Mais, de nos jours, les manifestations émeuvent assez peu ... Des youtubeurs publient une multitude de vidéos sensibilisant le grand public à cette question, les pétitions fleurissent, les interpellations prospèrent ... Et que fait M. Macron ? Il demande à un député de mon département, ancien avocat, qui fait mention sur LinkedIn de sa défense « d'une société pour concurrence déloyale et agissements délictueux dans le secteur du », de rédiger cette proposition de loi. Être député après avoir été avocat d'affaires n'est pas déshonorant, mais cela peut expliquer le déséquilibre manifeste du texte. Un texte soumis à un débat furtif, porté par un parlementaire trop peu soucieux de rassurer les inquiets, un calendrier couperet qui plane au-dessus de nos têtes, un texte dont on ne sait s'il bénéficiera aussi aux PME et aux start-up ou s'il vise les seuls grands groupes

Parmi ces amendements, je retiens une réponse faite à la lettre ouverte adressée lundi au Président de la République par d'innombrables lanceurs d'alertes, syndicats, associations, journalistes, chercheurs Dans cette lettre, signée notamment par la société des journalistes des et du deux titres dont on peut considérer qu'ils sont attachés au secret des affaires, tous ces citoyens demandent de restreindre le champ d'application de ce même secret aux seuls acteurs économiques concurrentiels. C'est le sens de l'amendement n° 51 rectifié du groupe socialiste. Monsieur le rapporteur, cela fait maintenant quelques années que nous nous croisons dans cet hémicycle. Je vous reconnais clarté et sincérité. Vous vous étiez opposé à la création du devoir de vigilance pour les sociétés mères, et votre action, respectable, de rapporteur va aujourd'hui d'abord vers le secret des affaires plutôt que vers un soutien à la liberté d'informer. Ce n'est pas vrai ! C'est en tout cas ainsi que j'interprète votre modification du texte initial supprimant le régime

Chers collègues, nous connaissons tous la force du symbole en politique. Ce matin, en commission des lois, François Pillet invitait le Sénat à se faire sentinelle des libertés publiques sur le projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Je partage son constat et appelle notre assemblée à faire de même avec les journalistes et les lanceurs d'alerte. M. Falciani, les syndicalistes du Bangladesh, les anonymes qui dénoncent parfois les comportements illégaux de leur entreprise, Mme Lucet- dont le travail n'est pas toujours prisé ici, au Sénat -sont autant de héros des temps modernes qui méritent sans aucun doute notre respect et notre protection. Il y a les héros de l'entrepreneuriat et de l'innovation il y a les héros de l'information et de la transparence. Ces derniers ne se retrouvent pas dans ce texte. Le Gouvernement et le rapporteur auront beau jeu de me répondre que ces héros se trompent et qu'ils ont mal compris cette initiative législative ; je ne partage pas cet avis. Et quand bien même je le partagerais, je jugerais utile de prendre notre temps

dans un contexte de compétition économique internationale toujours plus accrue pour les entreprises françaises, plusieurs initiatives législatives ont tenté, ces dernières années, de mettre en place, sans succès, un dispositif civil ou pénal de protection. Si le droit de la propriété industrielle est efficace pour assurer la protection des brevets, des marques et autres dessins et modèles, il n'est en revanche pas suffisant pour assurer celle des nombreuses informations économiques et techniques confidentielles des entreprises qui ne peuvent faire l'objet d'une protection juridique par un droit exclusif de propriété prévu par le code de la propriété intellectuelle. La transposition de la directive du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites permettra enfin à la France de se doter d'un tel régime de protection du patrimoine économique, technologique, de ses entreprises. Comme le prévoit l'article 19 de la directive, les États membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 9 juin 2018, l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer. Avant d'aborder le contenu de ce texte, je voudrais exprimer à cette tribune un regret- que je partage avec un grand nombre de mes collègues -quant au choix du Gouvernement de procéder à la transposition de la directive par une proposition de loi, à quelques semaines seulement de l'expiration du délai. Je ne Je ne peux que déplorer, en tant que législateur, l'examen en urgence et sans l'éclairage d'une étude d'impact de la transposition d'une directive de cette importance, à quelques semaines du terme du délai légal. Concernant le texte lui-même, je souhaite saluer les nombreuses modifications apportées par la commission des lois. En premier lieu, je me réjouis que la commission ait veillé à transposer plus fidèlement la directive et à clarifier les procédures judiciaires mises en place pour garantir une protection efficace du secret des affaires. Elle a ainsi renforcé la conformité du texte à la directive, en particulier sur la définition du détenteur légitime du secret, sur la caractérisation de l'obtention illicite du secret ou encore sur la portée juridique des exceptions au secret des affaires concernant les journalistes, les lanceurs d'alerte, ainsi que les représentants des salariés. Elle a également prévu que l'information protégée devait avoir une valeur économique, et pas seulement commerciale, pour couvrir des informations non protégées en l'état actuel, mais utiles pour une entreprise concurrente. Elle a renforcé la précision et la cohérence des procédures judiciaires mises en place par le texte, en particulier en matière de protection du secret des affaires devant les juridictions. Enfin, elle a veillé à la constitutionnalité du texte en supprimant l'amende civile spécifique prévue en cas de procédures abusives au titre du secret des affaires, jugée contraire au principe de proportionnalité des peines.

tout en clarifiant certaines des dispositions du texte. S'agissant des lanceurs d'alerte, elle a distingué plus clairement l'existence de deux régimes : l'un, issu de la directive, et l'autre, issu de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En effet, la transposition de la directive ne doit pas conduire à une remise en cause du régime français plus protecteur, En dernier lieu, dans le contexte de guerre économique auquel sont soumises les entreprises françaises par leurs concurrentes étrangères, je me réjouis que la commission ait créé un délit d'espionnage économique pour sanctionner le détournement d'une information protégée au titre du secret des affaires à des fins exclusivement économiques, excluant ainsi de son champ les journalistes, les lanceurs d'alerte et les représentants des salariés. Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, c'est avec la conviction de faire oeuvre utile en faveur de nos entreprises, exposées à une concurrence internationale de plus en plus importante, que le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi. La parole

Cette expression fait en elle-même l'objet de nombreux débats, interrogations, voire fantasmes ... Le droit français ne définit pas la notion de secret des affaires ; cette transposition représente, à n'en pas douter, une nouveauté juridique. Le code de commerce, même s'il mentionne le le secret des affaires dans les articles concernant la communication de certaines pièces, ne précise pas quelles informations doivent être protégées, selon quels critères, comment identifier le détenteur légitime et encore moins les exceptions au secret des affaires ni les procédures judiciaires pouvant être initiées à la suite d'une violation de ce même secret. Il est intéressant de noter également que la directive, dans sa version française, parle de « secret d'affaires » et non de « secret des affaires », comme le précise dans son très documenté rapport d'information notre collègue Philippe Bonnecarrère, remis au nom de la commission des affaires européennes. On constate souvent ce type de nuance dans la terminologie entre les instances européennes ou internationales et l'usage national. Je pense ainsi à la différence entre les droits humains et les droits de l'homme, dont il n'est pas toujours aisé d'évaluer les conséquences juridiques et pratiques. En outre, on associe souvent le secret des affaires à la culture et au droit anglo-saxons. Pourtant, on parle en anglais davantage de « », ce qui semble se rapprocher de la notion, bien française, de « secret commercial », voire de « secret industriel », à moins qu'il ne s'agisse ici encore d'un faux ami ... Ces terminologies mériteraient au moins d'être précisées, expliquées et explicitées. Il n'en reste pas moins que la présente proposition de loi vient combler un vide juridique, alors que sévit aujourd'hui une véritable guerre économique à l'échelle internationale

ou encore à l'affaire Volkswagen-General Motors, dans les années quatre-vingt-dix. Il y a une vingtaine d'années déjà, des agents de la CIA- ils ne s'en cachaient pas, au moins -pirataient des ordinateurs des institutions européennes afin de conforter les positions américaines lors des négociations du GATT. Plus récemment, une affaire de téléchargement illégal de données de l'équipementier automobile Valeo par une étudiante chinoise a défrayé la chronique. Toutefois, les affaires également récentes concernant certaines pratiques abusives, voire illégales, au sein d'entreprises ont vu l'émergence de nouveaux acteurs, comme les lanceurs d'alerte, aux côtés de la presse d'investigation traditionnelle. Depuis 2016 et la loi Sapin II, les lanceurs d'alerte bénéficient d'un statut juridique et d'une protection. Par ailleurs, la question de la responsabilité, notamment sociale et environnementale, des entreprises a été abordée lors du vote de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères. Enfin, le Parlement européen a connu de vifs débats, il y a deux ans, lors de l'examen de la directive sur la conciliation des notions de liberté et de protection. Tout l'enjeu est donc d'assurer un bon équilibre entre la liberté d'information au service de l'intérêt général et la nécessaire protection des connaissances à objet économique ou commercial, dans un monde qui nous interdit toute forme de naïveté. Je salue ainsi les garanties prévues pour la protection des journalistes, des syndicats ou des associations, dans le cadre des exceptions à la protection du secret des affaires. De même, la protection apportée au secret des affaires par la présente proposition de loi me semble essentielle, en particulier pour les PME, les TPE ou les start-up qui n'ont pas les moyens de lutter contre la captation de leurs secrets d'affaires. L'information protégée au titre du secret des affaires répondra ainsi à trois critères : son caractère non accessible non accessible de par sa nature ou sa conception, sa valeur économique effective ou potentielle et enfin le fait de faire l'objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. Le texte précise également les éléments d'appréciation à prendre en compte par le juge, notamment s'il y a lieu ou non de limiter la communication de certaines informations, la formation de jugement et les modalités de publication de la décision. La directive permet de rapprocher le cadre d'exercice de cette protection au niveau européen, mais demeure peut-être insuffisante, pour son application concrète, en ce qui concerne la coopération entre les États membres. Ainsi, des initiatives nationales qu'elle permet, allant jusqu'à la saisie de biens importés- s'ils sont issus d'un détournement de brevet ou d'un plagiat de modèle

Nous suivrons avec intérêt l'examen des articles et des amendements en séance. À cette heure, une large majorité des membres du RDSE est favorable au texte, avec les réserves déjà exprimées, tandis que quelques-uns s'y opposeront, faute de prise en compte de leurs amendements. La parole

ont signalé un vol d'informations confidentielles. Contrairement à la Chine, au Japon et aux États-Unis, l'Union européenne est l'un des derniers espaces économiques régionaux d'importance qui soit dépourvu d'une protection juridique harmonisée et d'une convergence juridique minimale en matière de protection des informations commerciales. Encore aujourd'hui, certains États membres de l'Union européenne ne disposent d'aucune protection des secrets d'affaires en droit interne, aussi surprenant que cela puisse paraître. C'est pour remédier à la fragmentation des législations nationales et à ce défaut de protection du développement de l'innovation que le Parlement européen et le Conseil ont adopté conjointement, le 8 juin 2016, la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués,

Avant de revenir plus en détail sur les principales avancées que porte cette proposition de transposition de la directive, permettez-moi de saluer le travail de la commission des lois, ainsi que celui de la commission des affaires européennes du Sénat, qui, dans le cadre de la procédure expérimentale, auront permis d'éviter des surtranspositions inutiles. Sur la forme, nous regrettons toutefois, comme la commission, le choix du Gouvernement de procéder à la transposition de la directive par une proposition de loi, nous privant ainsi de l'éclairage d'une étude d'impact. Par ailleurs, ce sont des délais d'examen excessivement contraints qui nous sont imposés, ce qui peut nuire à la qualité des débats parlementaires. Mais il s'agit là d'aspects formels. Sur le fond, le texte qui nous est proposé va indéniablement dans le bon sens, en permettant de protéger le patrimoine immatériel de nos start-up et de nos entreprises, en particulier les PME, qui disposent de moyens moindres pour lutter contre la captation de leurs secrets d'affaires. L'information protégée en tant que secret d'affaires se trouvera désormais clairement définie, de même que les cas d'obtention licite d'un secret d'affaires et, à l'inverse, les cas d'atteinte à ce dernier. Il en va de même des mesures susceptibles d'être prises par les autorités judiciaires, de l'octroi de dommages et intérêts et des mesures de protection du secret des affaires au cours des procédures judiciaires. Certaines marges de manoeuvre étaient laissées aux États membres, en leur accordant la possibilité, lors de la transposition, de prévoir une protection plus importante. Notre rapporteur, Christophe-André Frassa, a toutefois jugé que cette faculté n'était exploitée qu'a minima dans la proposition initiale et que les mécanismes civils mis en place en application de la directive étaient insuffisants. À l'aune de ces différents éléments, notre commission a apporté plusieurs modifications, afin d'aboutir à une transposition plus fidèle de la directive et de renforcer sa précision et sa cohérence. Il a tout d'abord été décidé de retenir une notion plus large de l'information protégée, en prenant en compte non plus uniquement sa valeur commerciale, mais aussi sa valeur économique. Nous avons également jugé bon de créer un délit de détournement d'une information économique protégée, dénommé délit d'espionnage économique. Ces peines complémentaires devraient être d'une portée plus dissuasive qu'une simple action civile et seront loin d'être inutiles dans un contexte international d'intense compétition économique. Par ailleurs, ce délit ne concernera que les personnes ayant contourné le secret des affaires afin d'en retirer un avantage de nature exclusivement économique. Dès lors, les journalistes, les lanceurs d'alerte et les représentants des salariés ne seront pas concernés. Ce sujet me conduit à aborder l'un des points centraux de ce texte, et l'une des principales difficultés : parvenir à la définition d'un juste équilibre entre la protection du secret des affaires et le respect des droits et libertés fondamentales. En effet, si les secrets d'une firme doivent indéniablement être protégés à des fins de compétitivité, ils ne sauraient servir à couvrir des pratiques répréhensibles et illégales, volontairement soustraites à la connaissance du public. Pour le dire autrement, la protection du secret des affaires ne saurait s'effectuer au détriment des consommateurs et de l'intérêt général. Des dérogations à la protection légitime du secret des affaires ont ainsi été prévues, et aucune procédure pour atteinte au secret des affaires ne sera recevable si ce secret est révélé au titre du droit à la à la liberté d'expression et d'information ou pour porter à la connaissance du public une faute ou une activité illégale. Par ailleurs, nous avons également veillé à ce que le régime français des lanceurs d'alerte, issu de la loi Sapin II, plus protecteur que celui issu de la directive, ne puisse pas être remis en cause. Seule ombre au tableau : la suppression, par notre commission, de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale introduisant un dispositif dit « anti-bâillons ». Il s'agissait, en créant une amende civile plafonnée, de prévenir les procédures abusives abusives que mènent parfois certaines entreprises en demandant des dommages et intérêts disproportionnés pour décourager les lanceurs d'alerte et entraver leur liberté d'expression. La commission des lois du Sénat a décidé de revenir sur cette disposition, pour des motifs d'inconstitutionnalité discutables, si l'on en croit notre collègue Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des affaires européennes. Nous suivrons toutefois l'avis de la commission des lois, en espérant que ces modifications ne porteront pas un trop grand préjudice aux lanceurs d'alerte. Mes chers collègues, parce que la transposition parce que la transposition de cette directive permet la mise en place d'un dispositif plus efficace de protection du secret des affaires pour les entreprises françaises et européennes, le groupe Union Centriste votera en sa faveur. La parole

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le Parlement a déjà eu, par le passé, plusieurs occasions de débattre de cette notion controversée de « secret des affaires ». Je ne rappellerai pas les multiples tentatives du député Bernard Carayon ni même l'amendement défendu, dans le même sens, par son collègue Richard Ferrand, à l'occasion de la discussion de la loi dite Macron. À la faveur d'une directive européenne votée en 2016, ce projet renaît par le biais d'une proposition de loi : curieux véhicule pour une transposition ! L'autre curiosité de ce texte réside dans les libertés que prennent ses rédacteurs avec le principe de subsidiarité. Le mécanisme de la transposition repose sur la volonté de remédier aux lacunes supposées du droit national par des dispositions qui l'enrichissent, le complètent ou le corrigent. En l'occurrence, plusieurs dispositions introduites par le texte de l'Assemblée nationale ont pour conséquence, d'amoindrir, voire d'abolir des avancées considérables du droit positif français ; je pense notamment au statut juridique du lanceur d'alerte. La Haute Assemblée veille, parfois avec un zèle excessif, à ce que les directives européennes ne fassent pas l'objet de transpositions excessives. En l'occurrence, il s'agit plutôt d'une sous-transposition et, pour certaines dispositions, d'une transposition régressive. On peut même se demander si l'absence d'étude d'impact et les imperfections juridiques nombreuses de ce texte ne sont pas destinées à cacher ce détournement manifeste de procédure. Il faut donc saluer favorablement l'initiative de la commission des lois, qui a restauré les droits des lanceurs d'alerte, tels qu'ils ont été définis par la loi du 9 décembre 2016. Protéger les lanceurs d'alerte, ce n'est pas, comme on le lit encore trop souvent, encourager la délation. C'est au contraire permettre aux individus d'exercer pleinement leur métier de citoyen, tel qu'il est défini dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, avaient alors considéré qu'il était du devoir des membres du corps social d'exercer leur « droit de réclamation », pour assurer « le maintien de la Constitution et le bonheur de tous ». Ce « droit de réclamation » est pour chaque membre de notre République une obligation aussi indispensable que celle qui impose, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, de donner avis au procureur de la République des crimes ou des délits dont il a connaissance. C'est l'instrument d'une démocratie rénovée pour laquelle chacun de ses membres agit en conscience pour la défense des intérêts collectifs. Il ne nous semble donc pas juste de confondre ces citoyens qui oeuvrent bénévolement et, parfois, malheureusement, au péril de leur situation familiale ou professionnelle et les pirates qui tentent de dérober des informations par fraude. C'est pourtant le risque que leur fait subir l'extension absolue du champ d'application de cette proposition de loi. La commission des lois du Sénat propose de créer, par un nouvel article du code pénal, un délit de détournement d'une information économique protégée. Il serait constitué à la condition que son auteur en retire un avantage de nature exclusivement économique. Il serait donc cohérent d'exclure du champ d'application de cette proposition de loi toutes les personnes qui agissent pour d'autres motifs qui sont visés par ce nouvel article du code pénal. En effet, considérer que toute divulgation d'information économique serait frauduleuse et qu'il reviendrait au donneur d'alerte d'apporter la preuve qu'elle ne l'est pas pourrait constituer une atteinte à l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sanctifie « la libre communication des pensées et des opinions Il nous semble donc indispensable de restreindre l'objet de cette proposition de loi aux seuls acteurs économiques et à ceux qui agissent pour eux. Cette redéfinition du champ d'application nous semble plus juste et plus efficace que le dispositif de la présente de la présente proposition de loi, qui mêle dans une même suspicion de principe tous les individus qui divulguent des informations à caractère économique, avant de consentir des dérogations que l'on sait, en droit, toujours incomplètes. Il eût été plus satisfaisant, au regard du devoir constitutionnel de réclamation, que le chercheur ou le journaliste, dans l'exercice de leurs missions, ne fussent pas contraints, pour agir, de prouver leur bonne foi devant les tribunaux et de subir parfois des procédures contentieuses dissuasives et des chicanes juridiques, dont l'unique objet est souvent de décourager tout débat contradictoire. Ainsi, dans sa rédaction actuelle, cette proposition de loi porte des dispositions qui ont pour conséquence d'amoindrir considérablement ou de neutraliser les avancées bénéfiques de la récente loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance En cela, il s'agit de nouveau d'une transposition régressive, et il eût été de meilleure politique que le Gouvernement assumât sa volonté politique de corriger ce texte et qu'il expliquât pourquoi cette loi, votée il y a tout juste un an, n'était pas satisfaisante. de loi, bricolée dans l'urgence et la précipitation, porte des objectifs bien éloignés de ceux de la directive dont elle prend prétexte, pour engager une refonte complète du droit positif récent sur le devoir de vigilance et le droit de réclamation. Enfin, nous restons dans l'attente d'une démonstration juridique solide de l'inadaptation de notre droit à protéger ce que vous appelez sans le définir de façon satisfaisante le secret des affaires. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion

Monsieur le président de la commission des lois, vous devriez demander aux services de faire l'inventaire de toutes les directives européennes qui n'ont pas encore été transposées, afin que, rapidement, une masse de propositions de loi émanant du Sénat

en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration de l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles

La protection a pour but de protéger contre la concurrence : elle ne doit pas nuire à la nécessaire transparence, notamment lorsque l'intérêt général est en jeu.

« rien dans la présente directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l'exercice de cette mobilité, la présente directive ne permet aucunement [ ...]

enfin le recours à la voie pénale. Le Conseil d'État lui-même dit : faites très attention à la voie pénale. La notion de secret des affaires est tellement floue que l'on ne sait pas comment elle peut être interprétée par des juges. Or on se précipite, monsieur le rapporteur, pour ajouter dans le texte de la commission une infraction pénale.

5, deuxième phrase : « Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement,

cette motion de renvoi à la commission changerait fondamentalement à la nature de nos travaux. Pour schématiser, nous suspendrions la séance

qui figuraient dans la directive pour les transposer. Vous avez en outre évoqué la question- nous nous la posons, bien entendu -de savoir si un certain nombre de scandales révélés récemment, notamment celui du Mediator,

Le scrutin est ouvert.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

nous pensons qu'il est essentiel que la protection contre la concurrence déloyale entre acteurs économiques, par ailleurs déjà réglementée par toute une série de dispositifs en droit positif- nous les avons déjà évoqués -, ne remette pas en cause les libertés fondamentales des citoyens ainsi que les compétences des autorités publiques en matière de droit à l'information. Or cet article est loin de répondre à cet impératif, tant dans la définition extensive qu'il propose du secret des affaires que dans les conséquences qui sont attachées à sa violation présumée. Cette proposition de loi, qui est marquée par un intense lobbying de nombreuses multinationales, illustre parfaitement le fait que le dialogue et la concertation ne sont pas toujours de mise dans le milieu des affaires. Pas d'étude d'impact- cela a été rappelé -, des auditions parfois confidentielles, menées rapidement, dans un délai contraint : à aucun moment le bien-fondé de ce texte n'a été vraiment démontré. La méthode ne convainc pas, et c'est assez justement que les journalistes, les lanceurs d'alerte et les ONG que nous avons réussi à rencontrer malgré ce délai contraint s'inquiètent fortement des conséquences de ce texte. Ils ne sont pas les seuls ! Ainsi, cela a été souligné, les acteurs de l'économie numérique, pourtant si chers à notre président, s'alarment aussi des risques pour l'innovation ouverte. En effet, le secret des affaires tel que défini à l'article 1

remis au Gouvernement, que le mot qui caractérise le mieux l'état d'esprit des Français sondés vis-à-vis des entreprises est malheureusement la méfiance. Ce texte ne fera que renforcer ce sentiment, l'opacité et l'irresponsabilité étant présentées comme les valeurs essentielles de l'entreprise. La protection de nos entreprises face à leurs concurrents internationaux soulève une

et protège des intérêts qui sont parfois opposés. C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi a reçu le soutien du Gouvernement. Je rappelle que toutes les informations qui sont détenues par les entreprises ne seront pas protégées ; seules le seront celles qui font l'objet de mesures raisonnables de protection à en conserver le caractère secret et qui ont une valeur commerciale effective ou potentielle. Cette protection accordée au secret des affaires ne signifie d'ailleurs pas qu'à l'avenir serait empêchée toute révélation dont

en particulier lorsqu'il s'agit de pratiques fiscales frauduleuses ou d'impact sur la santé et l'environnement, mais aussi l'intérêt des salariés. C'est donc une logique inverse qui devrait s'imposer, à savoir définir le cadre du secret des affaires là où il est légitime, c'est-à-dire dans le champ des acteurs économiques concurrentiels. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, que bon nombre d'amendements qui seront présentés à cet article, s'il n'était pas supprimé,

La mobilisation citoyenne autour du secret des affaires montre, s'il en était encore besoin, que sa protection apparaît comme une question particulièrement sensible, au carrefour de plusieurs droits et libertés fondamentaux. Pour cette raison, il est impératif que le champ d'application de la proposition de loi soit suffisamment délimité, afin que ce texte demeure un outil au service de la vie des affaires, sans possibilité de détournement, voire de contournement. Par cet amendement, nous souhaitons que les bénéficiaires de la protection du secret des affaires, les entreprises, soient explicitement mentionnés, comme vient de le dire ma collègue Marie-Noëlle Lienemann.

En effet, nous pensons, dans la droite ligne des travaux du Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, qu'il est nécessaire de rattacher le secret des affaires à la notion d'entreprise, afin de préciser l'objet de la proposition de loi ainsi que son champ d'application.

sans objet précis : les personnes morales de droit public, mais aussi des particuliers pourraient se prévaloir du secret des affaires. Or, sans étude d'impact, il est difficile de mesurer la portée d'une telle possibilité. À cet égard, les algorithmes pourraient tomber sous le coup de la protection du secret des affaires. Or les personnes publiques utilisent de plus en plus ce type d'outil. La mobilisation contre Parcoursup et de l'algorithme derrière APB nous rappelle, s'il en était besoin, la nécessité d'être particulièrement vigilantes et vigilants. Pour être acceptée et conserver une réelle efficacité, la protection des secrets d'affaires doit, comme son nom l'indique, conserver un certain ancrage dans la vie des affaires. Tel est le sens de notre amendement de précision. Quel est l'avis de la commission ? Cet

de la directive que nous devons transposer. En effet, une atteinte au secret des affaires peut émaner d'une personne qui n'est pas une entreprise sans pour autant être un journaliste, un syndicaliste ou un lanceur Si les atteintes au secret peuvent le plus souvent relever d'une concurrence déloyale entre entreprises confinant à ce qu'on appelle la « guerre économique »- c'est d'ailleurs la raison de la création par la commission du délit d'espionnage économique à l'article 1 -, elles elles peuvent aussi être le fait de personnes malveillantes qui ne sont pas des entreprises. L'avis de la commission sera donc défavorable pour tous les amendements de cette nature.

est fait mention de la « valeur économique, effective ou potentielle » de l'information protégée. Cela caractérise bien une information détenue par une entreprise. L'amendement est donc en quelque sorte satisfait. Au demeurant, la notion d'entreprise est matérielle et économique, et pas réellement juridique.

Selon le vocabulaire juridique de M. Cornu, peuvent être considérées comme « affaires » les « opérations de toute nature liées à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou financière C'est le sens de la première partie de notre amendement, qui tend à traduire cette définition dans le droit que nous sommes en train de constituer. Il s'agit dès lors de réserver la protection au titre du secret des affaires

Les informations protégées sont précisément définies, et l'atteinte à un tel secret ne peut être réparée que si sa divulgation porte gravement atteinte aux intérêts de l'entreprise victime. Ce dernier point fait écho aux recommandations de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen, qui a proposé de réserver le bénéfice de la protection aux seules informations dotées d'une « grande valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes et que leur divulgation porterait gravement atteinte à l'intérêt économique légitime de la personne qui en a licitement le contrôle », le contrôle », mais aussi à la proposition de loi Carayon, adoptée en 2012, qui prévoyait quant à elle que la divulgation non autorisée de ces informations doit être de nature à « compromettre gravement les intérêts de l'entreprise concernée en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux commerciaux ou financiers ». Cette définition permet donc de circonscrire précisément la notion de « secret des affaires », dans le respect de la directive européenne tout en protégeant véritablement les PME.

les quelques marges de manoeuvre offertes par la directive pour étendre plus encore la définition du secret des affaires. Parmi les critères auxquels doit répondre un secret des affaires, le texte retient le caractère connu ou accessible de l'information. Concrètement, la directive prévoit qu'une information relève du secret des affaires si elle n'est généralement pas connue des personnes appartenant au milieu qui s'occupe normalement du genre d'informations en question ou ne leur est pas aisément accessible. De ce point de vue, la transposition de ce critère par l'Assemblée nationale était, d'une d'une part, conforme à la directive et, d'autre part, satisfaisante sur le plan rédactionnel. M. le rapporteur a choisi de modifier ce critère pour retenir les « personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ». Derrière cette modification, présentée comme rédactionnelle, il y a en réalité une extension du critère : entre une personne qui agit dans un secteur ou un domaine d'activité s'occupant habituellement de cette catégorie d'informations et une personne familière de sites d'informations, il y a- vous l'avez noté -bien plus qu'une nuance Par ailleurs, et sur le plan de la rigueur juridique, il nous apparaît que la notion de personnes familières ouvre la voie à une abondante jurisprudence en raison de son flou ; « une personne agissant » nous apparaît une rédaction bien plus robuste et de nature à garantir la sécurité juridique à laquelle aspirent l'ensemble des acteurs.

c'est-à-dire « valeur commerciale, effective ou potentielle », puis « valeur économique » après le passage en commission. Si les autres éléments de la définition de l'information protégée ont une réalité assez directement accessible, ce n'est pas le cas sur ce point. Avec la notion de valeur économique, nous sommes par trop dans ce que j'appellerais « l'immatériel de l'immatériel », ce qui laisse la porte ouverte à bien des abus. C'est pourquoi nous proposons une définition plus précise reprenant la notion d'avantage concurrentiel, qui apparaît dès la première ligne du premier considérant de la directive, mais surtout dans une ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne, de 2016. la Cour précise que, vu sous l'angle de l'intérêt économique et commercial, le secret des affaires ne doit pas avoir une valeur en tant que tel ; il faut qu'il procure un avantage concurrentiel à son détenteur, de sorte que ce dernier ait un intérêt à le protéger. Il s'agit, dès lors, de protéger les informations qui constituent un avantage concurrentiel. Cela permet de mieux concilier protection du secret et liberté fondamentale.

la liberté d'informer et la divulgation d'informations dans un objectif d'intérêt général. En effet, cette définition très extensive de ce qui constitue une information protégée par le secret des affaires est problématique, d'autant plus que la commission a fait le choix de l'élargir encore, en parlant de « valeur économique ». Pour protéger les entreprises de la concurrence déloyale, tout en garantissant les libertés d'expression et d'information, il faut au contraire une définition plus stricte du secret des affaires, qui doit s'appliquer au champ concurrentiel uniquement et réguler les interactions entre les acteurs économiques. Tel est est l'esprit de cet amendement, qui vise à préciser la définition de l'information protégée comme ayant une valeur commerciale et conférant un avantage concurrentiel à l'entreprise du fait de son caractère secret.

ainsi que le prévoit l'article 2 de la directive. La commission des lois, sur l'initiative de son rapporteur, a substitué à la notion de « valeur commerciale » celle de « valeur économique ». Dans l'esprit du rapporteur, il existe de nombreuses informations que les entreprises veulent conserver secrètes alors même qu'elles n'ont pas de valeur commerciale, même potentielle, et dont la divulgation constituerait néanmoins une atteinte à l'entreprise. Certes, cette extension est autorisée par la directive, mais elle semble contraire à son esprit. Il existe sans doute des informations que les entreprises souhaitent conserver secrètes alors qu'elles n'ont pas de valeur commerciale, même potentielle ; simplement, si ces informations n'ont pas de valeur commerciale, elles n'ont pas vocation à être protégées au titre du secret des affaires. Elles pourront l'être au regard du code du travail, du droit pénal ou du droit de la responsabilité civile. Notre législation nous semble déjà suffisamment fournie pour ne pas laisser penser que les informations sans valeur commerciale, mais jugées stratégiques par l'entreprise, ne sont pas protégées.

52. Comme vient de l'expliquer notre collègue, nous souhaitons également rétablir la rédaction de la définition du secret des affaires telle que prévue dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, dans un souci de cohérence avec le droit européen et de rapprochement des termes utilisés dans la directive. Le considérant 14 de l'article 2 de la directive sur le secret des affaires prévoit explicitement qu'une information protégée par le secret des affaires revêt une valeur commerciale. Il précise par ailleurs certains critères qui déterminent la valeur commerciale, comme les intérêts économiques ou financiers, la position stratégique ou la capacité concurrentielle.

Je suis convaincue de l'absolue nécessité d'avoir une définition précise pour permettre la protection dans le strict cadre de ce que prévoit la directive. commerciale, effective ou potentielle, répond à ces exigences de précision et de fidélité par rapport au texte européen. Suggérée par le Conseil d'État dans son avis du 15 mars dernier, elle correspond à la lettre de l'article 2 de la directive tout en intégrant, comme je l'indiquais précédemment, les éléments d'interprétation qui figurent dans le considérant 14 de cette même directive. Cette expression permet ainsi d'englober le potentiel technique ou scientifique de l'entreprise, ses intérêts stratégiques ou concurrentiels, qui n'ont pas de valeur marchande. C'est pourquoi je propose de rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale.

C'est à l'entreprise de s'assurer que toute personne ayant accès à une information puisse en reconnaître facilement la nature confidentielle et ne puisse pas en faire usage ou la divulguer. La responsabilité de la protection de l'information doit lui revenir.

visant à restreindre le champ de la protection du secret des affaires aux seules entreprises et aux relations entre elles. la définition du secret des affaires qui est proposée n'est pas conforme à la directive que nous transposons.

il n'y a pas que les entreprises qui s'agressent et qui agressent ; il y a aussi des personnes malveillantes. Or restreindre à ce point le secret des affaires aux seules entreprises et penser qu'il n'y a qu'elles qui s'agressent ou se volent les secrets des affaires me

sans en modifier le sens. En effet, qu'est-ce qu'une « personne agissant dans un secteur d'activité »

je pense que vous en conviendrez avec moi. Je ne comprends pas comment la nouvelle rédaction adoptée par la commission étendrait le champ de la définition par rapport à la directive ni pourquoi elle serait plus floue que celle de l'Assemblée nationale, si vous me permettez une telle immodestie.

à revenir sur la modification adoptée par la commission, consistant à ce que l'information protégée par le secret ait une valeur économique et pas seulement commerciale, tout en exigeant le fait qu'elle confère un avantage concurrentiel à son détenteur. Sur ce second point, de nombreuses informations confidentielles ne confèrent pas nécessairement par elles-mêmes d'avantage concurrentiel à leur détenteur-

plus limitée, de « valeur commerciale ». La commission a voulu renforcer le niveau de protection en incluant des informations dépourvues de valeur commerciale en elles-mêmes, mais qui seraient utiles à une entreprise concurrente pour adapter sa propre stratégie.

innovantes dans la Tech -ou les informations stratégiques de l'entreprise encore confidentielles : projet de fusion ou de croissance externe, lancement d'un nouveau produit. Il s'agit effectivement d'une surtransposition ; je ne le cache pas. Elle est assumée comme telle et destinée à mieux protéger les entreprises françaises, comme le permet la directive. De plus, cette notion sera sans doute plus simple à apprécier pour le juge que celle de « valeur commerciale ». Au demeurant, le considérant 14 de la directive donne à la notion de valeur commerciale une interprétation tellement extensive qu'elle confine à la notion de valeur économique. La commission a donc émis un avis défavorable l'amendement n° 68 rectifié vise à rétablir une disposition supprimée par la commission, selon laquelle les mesures de protection raisonnable d'une information protégée pourraient « notamment

inutile, mais aussi source d'insécurité juridique pour les entreprises. Il n'est pas certain que la simple mention du caractère confidentiel d'une information pourrait toujours être jugée suffisante par un juge en tant que mesure de protection raisonnable. La commission a donc émis un avis

protection du secret des affaires plus étendue, sous réserve du respect de certaines dispositions impératives, notamment de la liberté d'expression. Il s'agit donc d'une directive d'harmonisation minimale. Cela signifie que les États membres ne peuvent pas, dans le cadre de la transposition, diminuer la protection

me paraît au contraire essentiel, pour des raisons de sécurité juridique au sein de l'Espace économique européen, que la définition du secret des affaires soit parfaitement harmonisée.

40 tend à rétablir le texte de l'Assemblée nationale, lequel prévoyait une stricte reproduction de la directive en vue de définir le caractère secret de l'information protégée. La rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat ne me paraît avoir aucune incidence sur le fond : je m'en remets donc à la sagesse

auteurs proposent en effet de préciser que cette valeur commerciale doit conférer un avantage concurrentiel à son détenteur.

effective ou potentielle, notamment lorsque l'atteinte qui est portée nuit au potentiel scientifique et technique, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle. L'adoption de ces amendements conduirait donc à méconnaître l'obligation de transposition de la directive.

dans un cadre précis. C'est ce qui rend le jeu juridique encore plus subtil, et je suis sûre que vous vous y livrerez avec grand plaisir. Vous l'avez évoqué, lorsqu'une directive est transposée,

semble assez réussi.

La question qui nous est posée est celle de l'extension de la définition du secret des affaires. Les uns pensent que la protection du secret des affaires doit s'arrêter aux informations qui touchent les intérêts commerciaux de l'entreprise. Les autres estiment, et c'est le cas de la commission, que la protection du secret des affaires doit concerner l'ensemble des informations économiques touchant l'entreprise.

avait pour objectif la protection des intérêts économiques français. Tout à fait ! Prenons des exemples très concrets. Une information sur la stratégie et les alliances d'une entreprise est économique, et non pas commerciale. Faut-il la protéger ou la livrer en pâture au public ? Une information sur le lancement à venir d'un nouveau produit révolutionnaire

Je réponds, avec la commission, assurément oui ! Il faut protéger toutes ces informations, et non pas avoir une conception restrictive du secret des affaires qui mette en péril l'intérêt de nos entreprises.

en date impliquant Facebook et Cambridge Analytica, qui ont récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d'utilisateurs. Nous serons tous d'accord pour indiquer que ni cette pratique ni les données recueillies ne constituent des savoir-faire qui légitiment une protection au titre du secret des affaires. En conséquence, cela va de soi, nous proposons de l'inscrire dans notre droit par la mention selon laquelle ne sont pas protégées au titre du secret des affaires les informations relatives à des données personnelles utilisées pour effectuer un profilage privé à des fins lucratives.

profilage commercial. D'une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d'être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l'entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles. D'autre part, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles et interdit de fonder des décisions sur la base exclusive d'un traitement de données de ce type, sauf lorsque ces traitements sont nécessaires à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat- cela vise en particulier le crédit et l'assurance -, sous le contrôle des autorités compétentes. Dans ces conditions, je ne je ne saisis pas très bien l'objectif recherché au travers de l'amendement : soit le traitement de données est conforme au RGPD, soit il ne l'est pas, mais dans tous les cas cela n'a pas grand-chose à voir avec la question du secret des affaires. En tout état de cause, le texte prévoit que le secret n'est pas

Gouvernement ? Le profilage est défini dans le RGPD comme une forme de traitement automatisé de données à caractère personnel qui consiste à utiliser ces données pour évaluer le profil de personnes physiques en matière de goûts, d'intérêts personnels, de santé, etc. Ces profilages peuvent être utilisés dans différents domaines, par exemple en matière de crédits, de mutuelles, de location de véhicules. Mais de telles pratiques sont rigoureusement encadrées, comme l'a dit M. le rapporteur, par l'article 22 du RGPD, qui interdit

En outre, la directive du 8 juin 2016 relative au secret des affaires prévoit elle-même l'articulation entre droit au respect de la vie privée et familiale, droit à la protection des données à caractère personnel Il en résulte que le secret des affaires peut couvrir les données à caractère personnel, mais uniquement si les droits de la personne concernée relatifs à ces données ne sont pas affectés. Autrement dit, le secret des affaires n'est pas opposable si les exigences du RGPD, telles que le droit à l'information, le droit d'accès, le droit de rectification,

pour notre part, que les données personnelles et leur traitement ne doivent pas avoir de valeur commerciale et ne peuvent pas être englobés dans le secret des affaires.

Pour qualifier les savoir-faire à protéger, la directive évoque tout à la fois la recherche et le développement, les investissements dans la production et l'utilisation du capital intellectuel, tout ce qu'on caractérise sous le mot d'« innovation Les esprits cyniques feront sans doute observer que les montages fiscaux de certaines entreprises traduisent une réelle capacité d'innovation. Quelle créativité, parfois ! Pour autant, il va de soi qu'ils ne constituent pas un savoir-faire à protéger au titre du secret des affaires. Nous jugeons indispensable de l'écrire explicitement dans notre droit. Enfin, je soulignerai que nous avons entendu l'observation du rapporteur sur le caractère trop imprécis de la notion d'optimisation fiscale. C'est pourquoi nous proposons d'exclure du champ du secret des affaires l'ensemble des mécanismes fiscaux mis en oeuvre par une entreprise.

de la protection au titre du secret des affaires les informations suivantes : l'impact environnemental de l'activité de l'entreprise, les conditions de travail de ses salariés, ses relations avec ses sous-traitants et ses filiales, les montages fiscaux-cela vient d'être évoqué -qu'elle peut avoir mis en oeuvre, ainsi que toutes informations permettant la prévention de la concurrence déloyale. Les entreprises ont besoin de pouvoir protéger les secrets les plus importants relatifs à leur politique commerciale ou à leur politique de recherche- c'est absolument incontestable. La vie des entreprises, du marché et de notre économie a besoin d'un minimum de secret. De même, il existe en France et en Europe des lois qui protègent le consommateur, par exemple sa sécurité et sa santé. Il Il ne s'agit pas de se battre contre l'entreprise, ni d'avoir une position caricaturale, mais bien de trouver un juste point d'équilibre. Aussi, la définition du secret qui nous est proposée n'est pas, selon nous, Le secret a besoin d'être encadré. Les précisions que nous apportons trouvent leurs origines dans l'actualité- il ne s'agit ni d'une vue de l'esprit ni d'une attitude dogmatique -, avec la multiplication de pratiques de management agressif, le recours excessif, voire illégal, aux contrats précaires, pollution de sites protégés, la sous-traitance inhumaine, la sous-traitance en cascade, qui permettent à de nombreuses entreprises d'échapper, dans de trop nombreux cas, à la plupart de leurs obligations. Les débats que nous avons eus sur la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard de leurs filiales et sous-traitants ont montré, si besoin était, l'ampleur des dégâts et la responsabilité des entreprises donneuses d'ordres. Nous pensons bien sûr, ici, aux travailleurs détachés ou aux révélations de certaines pratiques fiscales dites « dommageables ». On nous rétorquera que ces dispositions sont déjà couvertes par le droit positif. Nous répondons qu'il en est de même du secret des affaires. Cela ne nous empêche pourtant pas de légiférer aujourd'hui. Enfin, notre amendement s'inscrit dans un mouvement de fond, de réflexion, sur le droit des affaires, après l'émergence de la régulation et de nouveaux concepts, comme la conformité ou la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui sont aujourd'hui des notions phare pour promouvoir l'éthique des affaires. Quel

? L'amendement n° 48 tendait à soustraire les mécanismes d'optimisation fiscale de la protection du secret des affaires. Depuis la réunion, ce matin, de la commission des lois, cet amendement a été rectifié pour mentionner les mécanismes de nature fiscale élaborés par une entreprise, de sorte qu'on ne comprend plus très bien ce qui est visé. Qu'est-ce qu'un mécanisme de nature fiscale ? La rédaction, à mon sens, n'est pas très claire, alors même qu'elle ne l'était déjà pas ce matin ... Sur le fond, soit il s'agit d'optimisation fiscale licite,

ce qui est illicite, et là nous sommes dans le cas de la possible révélation par un lanceur d'alerte, car il s'agit de révéler une activité illégale. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. En tout état de cause, le secret des affaires n'est pas opposable à l'administration fiscale, laquelle peut d'ores et déjà procéder à tous les contrôles nécessaires et vérifier que ce qui est pratiqué est licite ou non. Le débat sur l'optimisation fiscale est,

Dans le même esprit, l'amendement n° 7 vise à soustraire de la protection du secret des affaires toute une série d'informations dans les domaines les plus variés, ce qui affaiblirait, à notre sens, singulièrement la protection des entreprises françaises et, surtout, ne serait guère conforme à la directive. Sur un certain nombre de points, cet amendement est satisfait, car le secret des affaires n'est opposable ni aux autorités administratives ou juridictionnelles dans leurs missions de contrôle ou de sanction ni aux lanceurs d'alerte qui divulguent des activités illégales ou des comportements répréhensibles : informations sanitaires ou environnementales, optimisation fiscale, fraude fiscale, infraction pénale ... L'avis est donc défavorable

à l'exclusion des mécanismes de nature fiscale élaborés par une entreprise, nous avons déjà vu qu'une information sera qualifiée de secret des affaires si elle réunit les trois critères qui sont précisés par la directive et que nous avons déjà évoqués. Cette directive ne prévoit pas la possibilité d'exclure par principe certains types d'informations de nature fiscale par exemple, ainsi que vous le proposez. En revanche, comme l'a relevé M. le rapporteur, un lanceur d'alerte qui signale un mécanisme d'optimisation fiscale pourra se prévaloir de la dérogation qui est prévue dans la proposition de loi que la directive institue à son profit, si le montage financier révélé peut être qualifié de comportement répréhensible. Ce sera le cas s'il porte atteinte à l'intérêt général. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. Je suis donc défavorable à cet amendement. L'avis est également sur l'amendement n° 7. Les auteurs de cet amendement expriment la crainte que, compte tenu de la protection accordée au secret des affaires, l'accès à certaines informations d'intérêt général ne soit plus possible, notamment dans le domaine de l'environnement, de la fiscalité, du droit du travail, de la lutte contre les fraudes, de la corruption. Je voudrais ici rassurer : il ne sera évidemment pas possible pour une entreprise de s'opposer aux enquêtes administratives ou judiciaires dont elle pourrait faire l'objet. Il ne saurait, là non plus, être question d'empêcher de révéler des fraudes fiscales, des manquements au droit du travail ou des actes de corruption sous quelque forme que ce soit. Cela est énoncé tout à fait clairement à l'article L. 151-6 du code de commerce. De plus, pourront être révélées les informations qui sont couvertes par le secret des affaires, lorsque cette révélation est faite dans le cadre de l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression et de communication ou encore dans le cadre d'un droit d'alerte. Je voudrais d'ailleurs répondre en

ce texte s'inscrit dans le cadre général de notre Constitution, laquelle porte à son plus haut point juridique la liberté d'expression, qui est donc la liberté première. Bien sûr, nous traitons ici d'un point singulier, mais tout cela s'inscrit dans un cadre constitutionnel. Je terminerai en disant que,

En effet, un certain nombre de choses sont en bordure, dans la zone grise. On ne peut donc pas considérer que ce sont deux choses totalement séparées. Cela étant, nous avons tout de même pris en compte vos remarques en commission, d'où notre tentative de trouver une formulation plus adaptée. Vous dites également que l'administration fiscale a les moyens. Elle dispose certes des moyens légaux du contrôle,

plus loin -de savoir-faire en matière d'optimisation fiscale, ce qui n'est pas illégal. La question est de savoir si l'optimisation fiscale

nous ne le confondons pas avec de la fraude fiscale, mais il est important que les responsables politiques, qui ont vocation à décider comment on lève l'impôt,

S'agissant des mécanismes fiscaux, il existe un point central : les prix de transfert. Les salariés devraient être en droit- c'est d'ailleurs le cas en Allemagne -de connaître l'établissement des prix de transfert. Je vous rappelle qu'une entreprise comme Colgate rapatrier en Suisse 90 % des profits qu'elle fait en France. Et après, on explique aux salariés qu'il faut qu'ils fassent des efforts, parce que leur entreprise n'est pas rentable ! Évidemment, on l'a dépouillée de sa rentabilité par les mécanismes de prix de transfert

Nous pensons que le texte de la proposition de loi, tel qu'il est rédigé, remet en cause l'intérêt général et le droit des citoyens à l'information. Il s'agit d'une inversion de nos principes républicains : le secret devient la règle et les libertés l'exception. De fait, en l'état, cette loi permettra de verrouiller l'information à la fois sur les pratiques et sur les produits commercialisés par les entreprises. Or de nombreux scandales sanitaires ou industriels récents démontrent la nécessité d'une transparence. Les entreprises ont aussi des responsabilités et doivent respecter le droit public à l'information, le droit de demander des comptes tel qu'énoncé par l'article XV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par cet amendement, nous souhaitons que la définition du secret des affaires pose le principe de la nullité des obligations de confidentialité dès lors qu'elles viseraient à faire obstacle à une révélation essentielle pour l'intérêt général. Quel

à la nature des produits mis sur le marché, ce qui entrave la bonne protection de la santé des citoyens et des citoyennes d'Europe. La réalité du moment, avant même cette directive, c'est une obstruction générale des grands groupes, notamment phytosanitaires,

malheureusement entravés dans leur travail de recherche par des groupes qui leur opposent de façon systématique le secret des affaires sur des informations qui touchent pourtant Je crains très sincèrement que le texte tel que vous voulez que nous le votions ne contribue à réaffirmer cette obstruction générale des grands

et républicain vise à reprendre une disposition de la directive selon laquelle l'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsqu'il est obtenu lors de l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. Sans cette précision, les représentants des salariés risqueraient régulièrement d'être mis en cause, notamment lors de la recherche d'un repreneur pour un établissement que l'entreprise mère souhaiterait fermer.

est parfaitement satisfait par les alinéas 35 et 36 du texte, auxquels je la renvoie et qui prévoient clairement une exception au secret des affaires pour l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés et de leurs représentants. Je sollicite donc le retrait de cet amendement, qui est, à mon sens,

sa créativité lorsqu'il a précédemment souhaité établir un distinguo entre le champ économique et le champ commercial et qu'il a fait appel au fait que le texte était en anglais. Il a sans doute oublié que le français était l'une des langues officielles de l'Union européenne

14, que chacun serait bien inspiré de relire, il indique très exactement : « Il importe d'établir une définition homogène du secret d'affaires sans imposer de restrictions quant à l'objet à protéger contre l'appropriation illicite. Cette définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques [ ...]. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. » Nous revenons sur ce point, qui a été

la protection d'informations sensibles. Traiter de l'usage illicite de ce qui est couvert par le secret des affaires devrait nous ramener à la question centrale du pillage technologique, l'espionnage industriel et de l'infiltration ne répondant le plus souvent qu'à un seul objectif : la concurrence économique dans ce qu'elle a de plus sauvage et de plus inadmissible. Nous ne vivons pas dans un monde de Bisounours ; parfois, tous les coups sont permis. Mais nous pensons tout de même que l'économie moderne ne fait pas obstacle au respect d'une éthique et de principes vertueux. L'espionnage industriel et le pillage des compétences et des savoir-faire aux fins de pratiquer une concurrence déloyale : voilà, selon nous, ce qu'il faut clairement combattre.

des informations obtenues, utilisées et divulguées par des entreprises qui profiteraient indûment des investissements réalisés par d'autres dans un contexte exclusivement concurrentiel, cela conformément à l'Accord sur les aspects La proposition de loi, telle qu'elle est actuellement rédigée, prévoit un dispositif de protection des savoir-faire et des informations commerciales. La nécessité n'en est pas contestée, mais il n'est pas mentionné que son champ d'application doit se restreindre au champ concurrentiel. En l'absence d'une mention limitant le champ de la protection du secret des affaires à l'exploitation déloyale dans le commerce, toute personne ayant un intérêt autre qu'économique à obtenir, à utiliser et à divulguer des informations protégées devra prouver qu'elle peut se prévaloir de l'une des dérogations

Ils seront ainsi dissuadés d'agir, ce qui porte préjudice à l'intérêt général. La liberté d'informer, la protection de l'intérêt général et des droits fondamentaux ne doivent pas être reléguées au rang d'exceptions au secret des affaires : il s'agit de principes fondamentaux.

tendent à limiter les cas dans lesquels l'obtention d'un secret est illicite à ceux où cette obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d'alerte ou les associations. En cela, ils ne sont d'ailleurs pas conformes à l'article 4 de la directive, qui n'est pas aussi restrictif. Le texte prévoit clairement Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes, les lanceurs d'alerte et les représentants des salariés- les auteurs des amendements n'ont d'ailleurs même pas évoqué ces derniers. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point. S'agissant des chercheurs,

il ne fallait pas restreindre la protection du secret des affaires aux seules relations entre entreprises. Des personnes autres que les entreprises peuvent porter atteinte au secret, sans pour autant être des journalistes, des lanceurs d'alerte ou des représentants des salariés. Pour ces raisons, l'avis de la commission est défavorable sur les quatre amendements. Quel

que le dispositif de protection du secret des affaires, tel qu'il est prévu et agencé par la directive et fidèlement transposé dans la proposition de loi, ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'une concurrence déloyale entre entreprises. L'obtention illicite d'un secret des affaires n'est pas toujours le fait d'une entreprise concurrente voulant tirer un profit illégitime de la connaissance qu'elle a ainsi acquise. L'obtention de l'information protégée peut un simple objectif de déstabilisation. Il peut aussi s'agir, comme vous l'avez précisé précédemment, monsieur le rapporteur, d'une action malveillante. En outre, ce n'est pas toujours non plus le fait d'une entreprise concurrente. Pour conclure, ainsi qu'on l'a dit à plusieurs reprises, il n'est juridiquement pas possible de restreindre la portée de l'article L. 151-3, compte tenu du niveau d'harmonisation prévu par la directive elle-même. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable sur les quatre amendements.

le rapporteur. Conformément à la définition des « biens en infraction » figurant à l'article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d'un secret des affaires la production, l'offre, la mise sur le marché, l'importation et l'exportation de produits résultant « de manière significative » d'une atteinte au secret- et non de produits résultant d'une atteinte significative au secret, rédaction qui anéantirait une partie de la protection prévue par la directive. Il procède également à deux coordinations

traduction du droit anglo-saxon, est étrangère au droit français et contraire à la jurisprudence constante de la bonne foi. En effet, pour la Cour de cassation, la mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés cette locution ruine donc la présomption de bonne foi et introduit un déséquilibre en droit français. Il convient d'inverser la charge de la preuve, en ajoutant, pour rétablir l'équilibre, la locution traduite du droit anglo-saxon « au-delà de tout doute raisonnable

est impossible. Les auteurs de ces amendements déplorent l'emploi du conditionnel, dans la formule « aurait dû savoir », en matière de connaissance du caractère illicite de l'obtention ou de l'utilisation d'un secret.

Gouvernement est également défavorable. Conformément au principe de droit commun relatif à la charge de la preuve, il appartient à celui qui se prétend victime d'une atteinte au secret des affaires de le prouver.

Le texte actuel de la proposition de loi engage la responsabilité d'une personne qui fait usage d'une information protégée au titre du secret des affaires, alors qu'elle sait ou aurait dû savoir que celle-ci a été obtenue ou divulguée de façon illégale. à défaut de pouvoir prouver que la personne qui a fait usage d'une information illicite savait que celle-ci avait été obtenue ou divulguée de façon illégale, on pourra présumer que cette personne aurait dû le savoir. Cette mention fait porter une suspicion sur l'intéressé, qu'il lui sera impossible de lever, d'autant que le texte n'impose aucune exigence concernant les modalités de la protection de l'information censée rester secrète. Or, si l'intéressé n'a pas eu connaissance du fait que l'usage de cette information relevait du recel, ce peut être aussi parce que l'entreprise n'a pas correctement protégé son secret. La défaillance d'une entreprise pourrait ainsi conduire à mettre en cause une

Gouvernement ? C'est à regret que j'émets un avis défavorable sur cet amendement. La rédaction proposée pour l'article L. 151-5 du code de commerce assure une transposition fidèle de la directive. Il ne me semble donc pas possible d'aller

prévoit que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires doit être considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national. Il est nécessaire de réserver également l'application des instruments internationaux dans cette hypothèse, en particulier les conventions bilatérales ou multilatérales relatives à la coopération judiciaire, comme la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves. Quel est l'avis de la commission ? Il s'agit d'une l'avis de la commission nous nous rapprochons de la loi de blocage, car cette convention encadre l'obtention des preuves dans un État étranger dans le cadre d'une procédure judiciaire. La commission est favorable à cet amendement.

M. Éric Gold. La commission des lois a modifié la rédaction des dispositions de l'article 1 concernant les exceptions à la protection du secret des affaires. Le texte adopté par la commission a ainsi substitué aux termes de « protection du secret des affaires » celui d'« opposabilité ». Cette modification nuit à l'intelligibilité des présentes dispositions. De plus, l'argument selon lequel cette rédaction serait davantage fidèle à l'article 5 de la directive du 8 juin 2016 ne semble pas convaincant, dans la mesure où cet article traite seulement des « dérogations » au secret des affaires. Il s'agit donc d'une interprétation du texte de la directive. Par cet amendement, nous proposons de rétablir la formulation retenue par l'Assemblée nationale, qui permet par ailleurs une plus grande protection des personnes visées par les exceptions à la protection du secret des affaires.

le secret des affaires n'est pas opposable, c'est-à-dire invocable lors d'une action en justice. Il prévoit en particulier que le secret des affaires n'est pas opposable dans le cadre de l'exercice du droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse et de la liberté d'information telle qu'établie par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. termes « y compris » qui posent problème à nos yeux. En effet, la protection de la liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des régimes démocratiques et, à ce titre, elle est garantie par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par ailleurs, comme cela est indiqué, la liberté d'information est garantie par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si l'inclusion de la liberté de la presse dans la liberté d'expression devrait aller de soi, le législateur a jusqu'à présent préféré la mentionner explicitement. Le choix des termes peut ainsi apparaître comme une restriction. Par ailleurs, cela nuit à l'intelligibilité de la loi. C'est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « y compris » par les mots « en particulier », afin de montrer qu'il s'agit d'une simple précision, concernant des principes qui doivent aller de soi.

droit à la liberté d'expression, de communication et d'information, telle qu'établie dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris le respect de la liberté de la presse.

n° 9. Il s'agit de faire en sorte que le secret des affaires ne puisse être invoqué de manière constante pour déclencher des procédures à l'endroit d'un certain nombre de personnes.

À la vérité, ce débat pourrait prendre une mauvaise tournure si nous retenions le pire pour ce qui est du droit des affaires et le pire pour le reste, c'est-à-dire la restriction des droits fondamentaux.

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. » On ne saurait être plus clair. La liberté académique, c'est le respect du travail des chercheurs scientifiques, qui ne sont pas soumis à une forme d'obligation de résultat et n'ont donc surtout pas de comptes à rendre au nom de je ne sais quelle logique commerciale et mercantile.

garde, nous priver de la possibilité de connaître des désordres sanitaires causés par certaines spécialités pharmaceutiques aux effets indésirables.

témoigne de l'importance accordée au sujet : « les entreprises comme les organismes de recherche non commerciaux investissent dans l'obtention, le développement et l'utilisation de savoir-faire et d'informations qui constituent la monnaie de l'économie de la connaissance et qui confèrent un avantage concurrentiel ». Les organismes de recherche, eu égard à leurs travaux en matière de développement et d'utilisation des savoir-faire, s'inscrivent sans débat possible dans le périmètre du secret des affaires. La question qui se pose au législateur est celle de l'articulation entre ces deux acteurs, car s'ils interviennent dans un même champ, ils n'oeuvrent pas au titre des mêmes intérêts, au point que, de plus en plus souvent, les chercheurs ou les enseignants-chercheurs font l'objet d'actions en justice en raison de leurs activités, celles-ci, d'intérêt public, pouvant entrer en contradiction avec les intérêts privés des entreprises.

ce matin en commission lorsque nous avons abordé l'examen de ces amendements : je ne vois pas pourquoi nous devrions instaurer un régime dérogatoire pour des enseignants-chercheurs qui, par principe, par fonction, par nature, ne sont pas

amendement. Monsieur le rapporteur, vous avez dit qu'il n'y avait aucune raison que les universitaires soient exclus

La rédaction de cet article élaborée par la commission des lois du Sénat distingue deux régimes de protection des lanceurs d'alerte, au risque de restreindre le champ d'application de l'exception. En revanche, la locution « y compris » figurant dans la rédaction de l'Assemblée nationale permet d'associer les deux définitions de manière cumulative, et ainsi d'assurer une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Par ailleurs, l'article 5 de la directive, d'application stricte, définit le lanceur d'alerte de manière plus large que l'article 6 de la loi de 2016.

Au nom du Gouvernement, je souhaite revenir au texte issu des travaux de cette assemblée. Je tiens d'abord à réaffirmer que l'article 5 de la directive définit plus largement le lanceur d'alerte que l'article 6 de la loi Sapin II, ce que traduisait justement la locution « y » figurant dans le texte voté par l'Assemblée nationale. Les lanceurs d'alerte au sens de la loi de 2016 bénéficient bien de la dérogation prévue par la directive.

renvoie non seulement à l'article 6 de la loi Sapin II, mais également à l'ensemble des dispositions de cette loi relatives au droit d'alerte. Cela induit que l'exception à la protection du secret des affaires ne serait effective qu'en cas de respect de la procédure d'alerte, condition qui n'est pas prévue par la directive, ce qui tend donc à restreindre le champ de l'exception.

La directive renvoie, notamment dans ses considérants et ses dérogations, à la complémentarité du droit de l'Union européenne et du droit national. Or la France a adopté le 23 mars 2017 la loi sur le devoir de vigilance, dont l'objet est de prévenir, autant que possible, « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement » résultant des activités économiques au sein des chaînes de valeur.

Le plan de vigilance est un instrument de garantie effective de droits fondamentaux, la valeur constitutionnelle des droits humains et des libertés fondamentales étant consacrée par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution

Labbé. Nous proposons de préciser que le secret des affaires n'est pas protégé dans le cas de la révélation d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général. Cet amendement vise ainsi à protéger les lanceurs d'alerte, notamment les personnes morales qui pourraient jouer ce rôle.

puissent bénéficier des mêmes exonérations que les personnes physiques lorsque l'intérêt général est en jeu. Les personnes morales, comme les ONG, ont tout leur rôle à jouer pour la protection de l'intérêt général.

Labbé. Cet amendement vise à concilier le secret des affaires et la loi sur le devoir de vigilance, adoptée le 23 mars 2017. Cela est permis par la directive, qui renvoie, notamment dans ses considérants et ses dérogations, à la complémentarité du droit de l'Union et du droit national. La loi sur le devoir de vigilance a pour objet de prévenir, autant que possible, « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement » résultant des activités économiques au sein des chaînes de valeur. Cette loi a représenté une avancée essentielle pour notre pays elle est d'ailleurs aujourd'hui reprise en grande partie par un groupe intergouvernemental de travail mandaté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le texte que nous examinons aujourd'hui ne doit pas permettre aux entreprises de réduire la portée de cette loi, notamment en matière de publication et de transparence,

le comprendra aisément, on ne peut que placer les lanceurs d'alerte en matière de fraude ou d'évasion fiscale hors du champ d'application du secret des affaires. Sans cela, nous n'aurions jamais eu vent des affaires Luxleaks, « Panama Papers » et autres, qui montrent à quel point certaines entreprises ont parfois pris de mauvaises habitudes en matière de fiscalité

objet de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale, qui faisait exception au secret des affaires dans le cas du signalement d'une faute, d'une activité illégale ou d'un comportement répréhensible, y compris pour l'exercice du droit d'alerte prévu par la loi Sapin II.

au moins dans l'attente de la directive annoncée sur les lanceurs d'alerte, et le dispositif de la loi Sapin II n'est en aucune manière remis en cause. Dans tous les cas, le problème de l'articulation entre les deux régimes demeurera, et la proposition de loi n'esquisse même pas un début de solution, la transposition de la directive se faisant vraiment sur cette question, par le recours à la locution « y compris », qui permet d'enchaîner l'un à l'autre. La rédaction adoptée par la commission est conforme à la directive, dès lors qu'elle préserve, dans toute sa pureté, le droit d'alerte général et inconditionnel prévu par l'article 5 de la directive. En tout état de cause, il était parfaitement inutile de mentionner dans ce texte le droit d'alerte inscrit dans la loi Sapin II, car le secret des affaires ne lui est pas opposable, ce qui ressort clairement de sa lecture. Le problème est même venu du fait que l'on veuille mentionner la loi Sapin II dans cette proposition de loi.

cette disposition ayant un objet limité aux conditions dans lesquelles s'applique l'exception prévue au bénéfice des lanceurs d'alerte en cas d'atteinte à un secret des affaires, elle n'aura pas d'incidence sur les mécanismes que les entreprises doivent mettre en oeuvre dans le cadre de leur devoir de vigilance, en application de la loi du 23 mars 2017. Ces mécanismes sont en effet autonomes. l'amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Labbé, l'alerte qui ouvre droit à une dérogation à la protection du secret des affaires peut porter sur une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. Cela signifie qu'elle peut être relative à des comportements qui, sans être illégaux, sont susceptibles de porter atteinte à l'intérêt général. Il ne fait ainsi aucun doute que les lanceurs d'alerte, au sens du droit interne,

est défavorable. Enfin, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 10, qui a pour objet d'indiquer expressément que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales autorise l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires. Il me semble que son adoption serait contre-productive, où elle nuirait à la bonne lisibilité de l'alinéa permettant aux lanceurs d'alerte de ne pas encourir de sanction pour avoir commis une atteinte au secret des affaires. Il est certain que l'objet de l'alerte peut concerner des faits de nature fiscale, et que leur révélation peut parfaitement contribuer à la lutte contre la fraude et

Le code du travail prévoit déjà un assujettissement au secret professionnel sur les procédés de fabrication, ainsi qu'une obligation de confidentialité sur les données par nature confidentielles en ce que leur divulgation pourrait nuire gravement aux intérêts de l'entreprise.

dans le cadre de « l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. » La Constitution prévoit un droit à la participation des travailleurs, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu'à la gestion des entreprises. L'utilisation et la divulgation aux salariés d'informations font partie intégrante des conditions permettant à ceux-ci de déterminer collectivement leurs conditions de travail, sachant que, par ailleurs, les élus sont toujours tenus, envers les salariés, à une obligation de discrétion issue du code du travail.

de manière générale, trois hypothèses d'atteinte au secret : l'obtention illicite, l'utilisation illicite et la divulgation illicite. Pour l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés et de leurs représentants, l'article 3 de la directive prévoit un cas d'obtention licite, pas d'utilisation ou de divulgation. Pour l'exercice légitime de leurs fonctions par les représentants des salariés, l'article 5 de la directive prévoit, lui, un cas de divulgation non illicite par un salarié, pas d'obtention ou d'utilisation, « pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ». Sur ces deux points, la proposition de loi est donc parfaitement conforme à la directive. L'avis de la commission est défavorable.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'insertion de dispositions concernant les relations de travail au sein du code de commerce n'est pas sans poser problème, surtout quand le code du travail comporte déjà des mesures suffisamment explicites en la matière.

Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées. » Par ailleurs, aux termes de l'article les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. par l'employeur. » Le code du travail comprend donc d'ores et déjà- vous vous en êtes préoccupée, madame la garde des sceaux, avec votre collègue la ministre du travail -des dispositions protectrices de la propriété industrielle et des savoir-faire propres à une entreprise et à sa production.

faisait du moindre bout de métal l'outil dont ses collègues tourneurs, fraiseurs, finisseurs ou polisseurs avaient besoin pour que leur production fût exactement comme ils l'entendaient. Cette culture-là n'a pas besoin de secret des affaires, juste de transmission. Elle reste la marque de fabrique de la classe ouvrière de notre pays. C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons, mes chers

revient au juge d'apprécier la responsabilité de ce salarié en fonction de son intention de divulguer le secret, dès lors qu'il ne relèvera pas des exceptions prévues au titre de la communication entre les salariés et leurs représentants ou de l'exercice du droit à l'information des salariés.

permette de citer l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux : « 1. Toute personne le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. « Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. « 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union. Au demeurant, le droit du travail encadre assez clairement les clauses d'exclusivité, dont il est quelque peu question ici, et il nous semble, dans l'absolu, que c'est au regard des règles fixées par le code du travail qu'il convient de prendre en compte le « secret des affaires Qu'on le veuille ou non, c'est aussi le savoir-faire des salariés, leurs compétences, leurs « tours de main » qui font la fortune d'une entreprise, aussi sûrement que l'engagement de ses actionnaires ou la pertinence de sa stratégie en matière de développement de la clientèle.

Il n'y a aucune raison que le dialogue naturel et normal entre salariés « de base » et représentants du personnel devienne un jeu d'énigmes parce que tout ne pourrait pas être dit.

En tout état de cause, les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité et au secret professionnel concernant les secrets dont ils peuvent avoir connaissance, indépendamment de toute clause de non-concurrence, sauf dans le cas des exceptions prévues par le texte en matière de communication avec les représentants des salariés. Pour cette raison,

ne pourrait avoir pour effet d'imposer aux salariés d'autres limitations que celles qui sont imposées par leur contrat de travail. Je rappelle qu'aucune disposition de la proposition de loi ne comporte de modification du droit du travail. Tel n'est d'ailleurs pas l'objet de la directive, ainsi

Les conditions dans lesquelles ces clauses peuvent être prévues entre un salarié et un employeur sont aujourd'hui très solidement fixées par une jurisprudence constante. Il n'est donc absolument pas justifié que la transposition de la directive conduise à remettre en cause l'état du droit sur ce point.

à donner compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions en responsabilité civile dès lors que les personnes poursuivies par une entreprise qui se considèrerait victime de la violation d'un secret des affaires s'adressent à un organe de presse.

texte expose ces acteurs à des procédures judiciaires pour prouver qu'ils se situent dans le cadre de dérogations au secret des affaires. Face à la presse, les juges des tribunaux de commerce

d'autant que les juges des tribunaux de commerce ne sont pas des magistrats professionnels : eux-mêmes issus du monde de l'entreprise, ils sont plus enclins à entendre les arguments des plaignants, quand ils ne sont pas tout simplement en plein conflit d'intérêts. Ce fut le cas

ainsi que des acteurs industriels majeurs qui sont favorables à ce que soit privilégiée la compétence des juges judiciaires des tribunaux de grande instance, sans pour autant que soit nécessairement retenue la compétence exclusive des juridictions parisiennes, comme c'est le cas en matière de brevets.

Le risque est grand que l'entreprise, afin d'obtenir une décision favorable, saisisse le tribunal de commerce de cette violation, en agissant non contre le journaliste, mais contre l'organe de presse, société de droit privé.

D'une part, la possibilité pour le juge de prendre seul connaissance d'une pièce couverte par le secret des affaires devient un préalable systématique à tout aménagement du principe de contradiction. Or il me semble préférable de laisser au juge toute latitude pour décider de la mesure la plus adaptée en vue de protéger le secret dans le respect des principes fondamentaux de la procédure civile, ainsi que le prévoyait le texte issu de l'Assemblée nationale. D'autre part, est supprimée la faculté offerte au juge de ne communiquer la pièce litigieuse qu'aux seuls avocats des parties. Cette possibilité est importante en pratique, particulier lorsque le juge a besoin d'être éclairé d'un point de vue technique sur la pertinence d'une pièce pour la solution du litige et qu'il ordonne une expertise à laquelle seuls les avocats peuvent assister. Elle protège efficacement le secret des affaires puisque, en application de l'article L.153-2, l'avocat est soumis à une obligation de confidentialité à l'égard de son client. Cette mesure est autorisée par le paragraphe 2 de l'article 9 de la directive, qui est d'harmonisation minimale. Elle est strictement encadrée. Le juge ne peut envisager de limiter la communication d'une pièce aux seuls avocats que si la protection du secret des affaires ne peut être autrement assurée et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense. Il ne pourra jamais y recourir si la pièce est nécessaire à la solution du litige.

Il ne fait aucun doute que l'obligation de confidentialité issue du premier paragraphe de l'article 9 de la directive est applicable à toute personne morale partie à une procédure prise en la personne de son représentant légal ou statutaire. Toutefois, la commission des lois s'est interrogée sur les modalités de l'application de cette obligation de confidentialité aux personnes morales et elle a proposé une modification de l'article L.153-2 qui ne me semble pas conforme à l'esprit de la directive. Je propose donc de clarifier cette disposition. D'une part, il sera précisé que, lorsqu'une partie est une personne morale, l'obligation de confidentialité s'applique tant à ses représentants légaux ou statutaires qu'aux personnes qui la représentent au cours de l'instance et qui peuvent être, par exemple, des salariés. D'autre part, je propose de rétablir le troisième alinéa de l'article L.153-2 dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, afin d'expliciter le fait que l'obligation de non-confidentialité n'est pas applicable entre la personne physique qui représente la personne morale lors de l'instance et les représentants légaux ou statutaires de cette personne morale. Dans la mesure où un salarié peut représenter devant la juridiction la société dans laquelle il travaille, il devra rendre compte des débats auprès de son employeur, du représentant légal ou statutaire de cette société. Dans cette situation, il ne peut en effet y avoir application d'une obligation de confidentialité entre le salarié et l'employeur puisque le principe du contradictoire s'apprécie en la personne représentante légale ou statutaire de la société partie à la procédure.

et 32 rectifié visent à réserver au seul tribunal de grande instance, voire au seul tribunal de grande instance de Paris, la compétence pour connaître des actions relatives aux atteintes au secret des affaires. En application des règles normales de compétence juridictionnelle, le tribunal de commerce sera compétent en cas de conflit entre deux entreprises concurrentes- commerçants ou sociétés commerciales, y compris sociétés de presse. C'est

insupportable. Quoi que chacun puisse penser du tribunal de commerce, celui-ci ne pourra pas connaître d'une affaire mettant en cause un journaliste, un lanceur d'alerte, un syndicat ou une association.

Comme les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce devront appliquer la loi, éclairés par la jurisprudence des cours d'appel et de la Cour de cassation, dans le respect des principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité des juridictions, sans préjudice des voies de recours pour les personnes condamnées.

la systématisation des mesures de protection du secret des affaires lors de toutes les procédures judiciaires est un apport important de l'Assemblée nationale. Or les auteurs de cet amendement prétendent que ces dispositions ne sont pas utiles, car elles seraient déjà satisfaites par l'ordonnance du 9 mars 2017 concernant la réparation des dommages résultant d'une pratique anticoncurrentielle. Ce n'est pas exact. En effet, les mesures mises en place par cette ordonnance ne concernent que les actions en matière de dommages de concurrence, et non pas toutes les actions judiciaires pour lesquelles une question de protection du secret des affaires peut être soulevée. L'article 1 de la proposition de loi supprime d'ailleurs ces dispositions spécifiques en matière de concurrence au profit de ces nouvelles dispositions générales.

texte de l'Assemblée nationale, alors que celui-ci n'est pas tout à fait conforme à l'article 9 de la directive s'agissant des mesures que le juge peut prendre pour préserver le secret des affaires d'une pièce discutée dans la procédure.

Pour autant, adopter cet amendement porterait une atteinte forte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, ce qui a justifié la décision de la commission d'en rester aux préconisations de la directive. Ainsi, l'article 9 de la directive ne permet pas au juge de prendre seul connaissance de la pièce sans aucune forme de communication aux parties. Dans le texte de la commission, il s'agit bien d'une prise de connaissance préalable par le juge, effectivement systématique lorsqu'une partie invoque le secret pour une pièce afin de voir s'il y a lieu ou non de prévoir des mesures particulières de protection pour cette pièce. En tout cas, ce n'est pas une mesure de protection en soi, car il y a de de toute façon, ensuite, une communication aux parties. Sur ce point, le texte de l'Assemblée nationale a été contesté avec constance lors de toutes les auditions, que ce soit par les professionnels, par les magistrats ou par les avocats. L'article 9 de la directive ne permet pas davantage de limiter l'accès d'une pièce aux seuls avocats des parties, même si cela a été présenté lors des auditions comme une piste intéressante. La directive exige l'accès d'au moins une personne et un avocat pour chaque partie. C'est ce que prévoit le texte de la commission. Sur ce point, peut-être pourrions-nous envisager une limitation aux seuls avocats des parties, mais, de toute façon, le texte prévoit une obligation de confidentialité pour toutes les personnes ayant accès à la pièce. Pour toutes

à la procédure. Les personnes représentant la société devant le tribunal étaient tenues à l'obligation de confidentialité, mais non envers les dirigeants de la société, lesquels n'étaient soumis à aucune obligation de cette conduisait immanquablement à la fuite par le haut du secret des affaires. Pour remédier à cette incohérence, la commission a prévu une obligation de confidentialité à l'égard des dirigeants de la société. L'amendement n° 63 du Gouvernement

pour objet une atteinte au secret des affaires. Je ne crois pas justifié de déroger, pour ces actions, aux règles de droit commun, qui attribuent compétence au tribunal de commerce pour les contestations entre commerçants, entre sociétés ou relatives aux actes de commerce. S'agissant des actions qui pourraient être engagées contre des journalistes ou des particuliers non commerçants pouvant répondre à la définition du lanceur d'alerte, je rappelle qu'elles ne pourront être introduites que devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. C'est une logique juridique ; il ne me semble donc pas utile de le préciser.